La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 15 février 2024 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n’y a pas d’observation ?… Le procès verbal est adopté.

portant respectivement sur les articles 1, 2 et 4 de la proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien être des femmes au travail, Patricia Schillinger souhaitait voter pour.

Acte est donné de ces mises au point, mes chers collègues. Elles figureront dans l’analyse politique des scrutins concernés. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai l’honneur de vous présenter ce projet de loi organique, dont est simple, puisqu’il prévoit le report des élections provinciales de Nouvelle Calédonie à une date non fixée, mais ne pouvant aller au delà du 15 décembre de cette année.

Cette déconnexion croissante entre le corps électoral spécial et le corps électoral général est un sujet politique majeur

On peut admettre qu’au nom de la citoyenneté calédonienne le droit de vote pour les élections provinciales soit restreint aux personnes solidement établies sur le territoire autonome de Nouvelle Calédonie. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement ne vient pas vous demander de dégeler totalement le corps électoral pour les élections provinciales ; il accepte l’idée

C’est donc avec la modération nécessaire que le Gouvernement, qui entend la préoccupation politique, symbolique et bien sûr électorale de chacun des partis politiques qui composent la Nouvelle Calédonie et qui sont reconnus par la Constitution comme concourant à la démocratie, qu’après trois référendums d’autodétermination ayant conclu au maintien sans contestation de la Nouvelle Calédonie dans la République française, il n’est plus acceptable, d’un point

! – et de voir des Calédoniens nés en Calédonie ne pas pouvoir voter à des élections locales. Dans ce contexte, le Gouvernement, puis le Chef de l’État lui même à Nouméa,

Le gel du corps électoral n’est conforme ni aux principes essentiels de la démocratie ni aux valeurs de la République. C’est une position politique que l’État assume depuis très longtemps et pas seulement une préoccupation d’ordre juridique. la vie démocratique et la continuité des institutions ne peuvent s’interrompre éternellement faute d’un accord local. Il ne s’agit pas pour le Gouvernement de changer la façon dont les électeurs pourraient choisir leur avenir institutionnel.

Techniquement, l’État est en mesure de tenir cette échéance. Le projet de décret pour réviser les listes électorales est prêt. Il est même dans mon dossier et à votre disposition.

des emplois par milliers. Je rappelle que le gouvernement autonome de Nouvelle Calédonie gère les sujets sociaux. En d’autres termes, c’est par les cotisations payées par les Calédoniens eux mêmes

Le Gouvernement de la République n’a pas ménagé ses efforts pour créer les conditions d’une négociation entre toutes les parties depuis la convention des partenaires au mois de novembre 2022. Nous ne pouvons que nous féliciter qu’un dialogue local entre les deux camps ait enfin pu s’établir, comme le démontre le communiqué de presse de l’ensemble des parties publié voilà plusieurs semaines.

qui ont su, dans l’histoire de la République, trouver entre eux des accords leur permettant de construire le présent et l’avenir du territoire.

qu’il faut organiser et que l’on ne peut pas suspendre et, de l’autre, l’avenir de la Nouvelle Calédonie. Sur la démocratie calédonienne dont nous avons à débattre, le texte paraît simple : il s’agit de reporter les élections.

initiale. Alors même que le processus juridique de transition qui a été amorcé par l’accord de Nouméa et organisé en application de cet accord par une révision constitutionnelle est achevé, pose évidemment problème. Je ne discuterai pas ici du problème de principe : après tout, dans le passé, on a admis que les Calédoniens, par un accord passé entre eux, puissent proposer des dérogations à l’égalité de suffrage.

Quoi que l’on pense des arrangements qui ont été trouvés dans le passé et de leur devenir, il faut bien que des élections soient organisées. Si elles l’étaient sur le fondement de la liste actuelle,

supplétif un projet de loi constitutionnelle visant à modifier la liste électorale, de sorte que celle ci puisse se rapprocher de l’inscription de l’ensemble des Français en âge de voter, sans tout à fait atteindre ce périmètre. Aussi, pour que l’on ait le temps soit d’adopter une révision constitutionnelle, soit de permettre la conclusion d’un accord qui serait ensuite traduit par des textes constitutionnel et organique, il est nécessaire de reporter les élections. Ce n’est tout de même pas une bien grande affaire que de reporter les élections dans une collectivité territoriale ! Nous avons de nombreux précédents, qui ont permis au Conseil constitutionnel de définir les conditions

que la durée de la prolongation soit raisonnable. Une discussion a eu lieu à ce propos. Après tout, le ministre est chef de son administration et, s’il nous assure que son administration est capable d’organiser un scrutin d’ici au 15 décembre prochain

le Gouvernement n’évince pas le Parlement, qui trouve un intérêt à soutenir ses démarches dans la mesure où il peut ainsi en vérifier le bien fondé.

au motif d’intérêt général du report des élections est remplie, puisque l’on ne peut pas organiser ces dernières sur les bases actuelles, d’autre part, que la date du 15 décembre n’est pas trop éloignée.

ministre, forts d’une longue expérience d’évolutions de la Nouvelle Calédonie décidées par la négociation entre les Calédoniens sous l’égide de l’État, l’État, nous continuons de préférer cette formule. C’est pourquoi j’ai qualifié la révision constitutionnelle, sans faire offense à notre loi fondamentale, de « méthode supplétive

avancer sur le fondement d’un consensus plutôt qu’en nous appuyant sur une démarche que vous avez vous même qualifiée d’« unilatérale » et qui ne peut constituer que la dernière option, à défaut de toutes les autres. Voilà ce que je tenais à vous dire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a maintenant plus de trente cinq ans, la Nouvelle Calédonie était au bord de la guerre civile. Michel Rocard, alors Premier ministre, et Louis Le Pensec, alors ministre des départements devaient relever des défis majeurs : ramener la paix, renouer les liens de la confiance et engager un mouvement de décolonisation pacifique et viable. Les accords de Matignon en 1988, puis l’accord de Nouméa en 1998 ont été de grands tournants pour maintenir la paix civile après le drame d’Ouvéa, puis l’assassinat de Jean Marie Tjibaou. Si la situation avait atteint un tel paroxysme, c’est en partie à cause de la marginalisation politique et économique des Kanaks, mais aussi, et surtout, en raison des manquements à la parole donnée par la France. En 2008, dans une tribune commune, Michel Rocard et Lionel Jospin écrivaient : « Au terme du processus, entre quinze et vingt ans après la signature de l’accord de Nouméa, soit entre 2014 et 2018, la Nouvelle Calédonie disposera donc de la quasi totalité des compétences et des attributs de la souveraineté, ses citoyens seront appelés à se prononcer pour savoir s’ils souhaitent le transfert des dernières compétences exercées par l’État. Cette construction originale doit permettre de bâtir un destin commun pour cette population pluriethnique, constituée du peuple d’origine et de ceux qui, depuis un siècle et demi, s’y sont installés durablement. Ce destin commun s’affirmera, soit dans la République française, soit dans un pays dont les liens avec la France seront à définir. » Le processus engagé par l’accord de Nouméa et les trois consultations portant sur l’accession à la pleine souveraineté sont arrivés à leur terme le 12 décembre 2021, même si la troisième consultation pose de nombreux problèmes en termes d’organisation, de participation et donc de légitimité. Le Gouvernement s’est entêté à maintenir cette troisième consultation, sortant alors de sa neutralité et provoquant ainsi une période de blocage. Il est clair que les élections les élections provinciales qui doivent se dérouler entre le 12 avril et le 12 mai 2024 ne peuvent pas avoir lieu avec les listes électorales actuelles, qui excluent de trop nombreux Calédoniens.

Dès lors, nous approuvons dans son principe le report des élections et nous proposerons même la date du 30 novembre 2025 au lieu du 15 décembre 2024. Il s’agirait alors d’un report de dix huit mois, une telle durée, acceptable selon l’avis du Conseil d’État, nous semblant beaucoup plus adaptée pour laisser du temps aux discussions en cours. cours. En effet, le consensus politique doit être la priorité absolue. Un accord global entre les parties doit être trouvé, afin de permettre à la Nouvelle Calédonie de disposer d’un cadre institutionnel stable au cours des prochaines décennies.

de la rencontre entre les loyalistes et les indépendantistes à Bourail et grâce à la démarche constructive de l’UNI Palika. C’est une bonne nouvelle, car le dialogue demeure le seul chemin viable pour parvenir à un accord politique pérenne. tenu de la reprise du dialogue, nous ne comprenons pas la pression qu’exerce le Gouvernement en liant le présent projet de loi organique à un projet de loi constitutionnelle, qui sera examiné dans quelques semaines et risque de compromettre les discussions en cours. Nous proposerons également un amendement visant à réaffirmer l’impartialité et le rôle moteur de l’État dans les discussions. Rappelons ici que la nomination au Gouvernement de Sonia Backès fut un très mauvais signal. De plus, présenter un projet de loi partiel, ayant pour seul objet l’élargissement du corps électoral, risque de compromettre toutes les chances d’aboutir à un accord global et de cristalliser les antagonismes. je citerai de nouveau les mots de Michel Rocard et de Lionel Jospin : « Plus que jamais, il faut parler, diagnostiquer sans complaisance les injustices qui persistent et y porter remède, rechercher ce qui rassemble et discuter ce qui divise. L’État, partenaire politique des accords, en charge de l’avenir de la Nouvelle Calédonie, doit assurer une mission permanente de dialogue. Il ne doit pas relâcher ses efforts et sa vigilance. […] La question calédonienne est d’intérêt national.

Il vise à reporter au plus tard au 15 décembre 2024 les élections des membres du congrès et des assemblées de province en Nouvelle Calédonie. Nous aurions certes préféré respecter le calendrier électoral initial. Ces élections auraient dû en effet se tenir dans moins de trois mois, soit au mois de mai prochain. Néanmoins, la réalité de la situation politique calédonienne nous impose ce report pour que ces élections respectent des exigences démocratiques fondamentales.

Cela a été dit, plus de 42 000 électeurs calédoniens sont aujourd’hui exclus du corps électoral provincial, sur un total de 221 000 électeurs.

Vous admettrez que cette situation serait inacceptable au regard des exigences démocratiques de notre République ! Parmi ces 42 000 citoyens français ainsi privés du droit de vote aux élections provinciales,

en faire partie. La prolongation de sept mois, soit jusqu’à la fin de cette année, du mandat des assemblées actuelles vise donc à nous laisser suffisamment de temps pour réviser la Constitution et mettre fin au gel du corps électoral provincial. Certains partis indépendantistes approuvent également ce report. Consulté sur ce projet de loi organique, le congrès de la Nouvelle Calédonie a émis, à une large majorité, un avis favorable. Les Calédoniens, dans leur très grande majorité, veulent que les assemblées locales soient renouvelées sans tarder, afin de renforcer leur légitimité démocratique. C’est pourquoi je serai opposé à l’amendement déposé par nos collègues socialistes, qui vise à reporter les élections provinciales jusqu’en novembre 2025. Depuis mai 2019, la Nouvelle Calédonie vit une situation politique paradoxale. Elle est dirigée au congrès et au gouvernement par une majorité indépendantiste, alors même que, à trois reprises – en 2018, en 2020 et en 2021 –, lors des consultations référendaires d’autodétermination, les Calédoniens se sont largement exprimés en faveur du maintien de la Nouvelle Calédonie dans la République. République. La détérioration économique particulièrement grave que connaît notre territoire, au regard notamment de la situation de sa filière nickel, impose des décisions fortes qui ne peuvent être prises que par des assemblées relégitimées par le suffrage universel des Calédoniens. Il est donc urgent, monsieur le ministre, que se tiennent de nouveau des élections et que le délai maximal du 15 décembre 2024 soit tenu. faut, mes chers collègues, prendre la mesure de l’importance d’un report de ces élections. Je vous invite donc à accueillir favorablement ce projet de loi organique, indispensable pour la Nouvelle Calédonie, dans la version qui nous est proposée par la commission et à l’adopter avec la majorité la plus large possible. La

De par son statut particulier, elle dispose d’un partage de souveraineté avec l’État, bien que cette notion fasse l’objet d’un débat doctrinal parmi les juristes. Elle bénéficie de ses propres institutions : un congrès, un sénat coutumier et Elle jouit aussi d’une autonomie partielle et peut ainsi voter des lois du pays dans certains domaines énumérés par la loi organique qui détermine son statut. Cette année 2024 est particulièrement importante pour la Nouvelle Calédonie. En effet, deux projets de loi lui seront projet de loi constitutionnelle visant à modifier le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province, qui sera examiné au mois de mars au Sénat, et un projet de loi organique visant à reporter les élections de ces mêmes institutions. Je ne m’attarderai pas sur le premier projet de loi, dont nous aurons l’occasion de débattre pleinement dans cet hémicycle dans quelques semaines. J’espère encore qu’un accord pourra être trouvé entre les acteurs politiques locaux, dans l’intérêt de tous les Calédoniens et, plus largement, de notre démocratie. Le second projet de loi porte sur les élections qui devaient se tenir en mai prochain. Il vise à les reporter au plus tard au 15 décembre de cette année. Avec le texte

Sur ce point, le fait est qu’il n’apparaît plus légitime aujourd’hui de procéder à des élections en Nouvelle Calédonie sans réinterroger au préalable la composition du corps électoral. Je le rappelle, celui ci a été restreint en 1998 à la suite de l’accord de Nouméa. Le corps électoral a ensuite été tout bonnement gelé lors de la révision constitutionnelle de 2007. de 2007. En 1998, nous étions tout juste dix ans après le drame d’Ouvéa. Vingt cinq ans plus tard, le contexte et l’évolution démographique nous éloignent encore davantage de ce qui avait alors justifié une dérogation à certains principes constitutionnels. Surtout, les conditions fixées par l’accord de Nouméa et qui devaient conduire à réinterroger la composition du corps électoral ont été satisfaites. Je pense notamment aux trois référendums sur l’indépendance de la Nouvelle Calédonie qui ont eu lieu en 2018, Il est donc désormais nécessaire et légitime d’avoir ce débat, lequel devra cette année trouver une issue afin que les élections puissent se tenir. Reporter les élections en 2025 ne me semble pas raisonnable.

J’espère que, avec ce report et le projet de loi constitutionnelle que nous examinerons au mois de mars, nous pourrons leur apporter rapidement des réponses afin que la Nouvelle Calédonie puisse avancer dans la sérénité et dans l’unité. Elle en a bien besoin.

par les accords de Matignon du 26 juin et du 20 août 1988 et l’accord de Nouméa du 5 mai 1998, la Nouvelle Calédonie s’est engagée dans un processus unique, négocié et ensuite constitutionnalisé, d’émancipation au sein de la République française. Depuis de nombreuses années, la Chambre haute a multiplié les initiatives pour permettre un suivi attentif du dossier calédonien : création d’une mission d’information dont j’ai eu l’honneur d’être l’un des rapporteurs ; mise en place d’un groupe de contact spécifique présidé par le président du Sénat, Gérard Larcher cela témoigne de l’importance, comme l’a rappelé le rapporteur, que nous attachons au sujet – ; nombreux rendez vous avec les autorités et les groupes politiques calédoniens. Nous sommes arrivés aujourd’hui au bout du chemin engagé il y a trente cinq ans. Les Calédoniens ont choisi de demeurer au sein de la République à trois reprises. Toutefois, nous devons noter que l’expression d’une majorité s’est érodée au fil des consultations et que le troisième référendum a fait l’objet d’une abstention massive, à hauteur de 56 % du corps électoral, le FLNKS ayant décidé de ne pas y participer. Eu égard à l’histoire du pays, d’une part, et aux résultats des consultations d’autodétermination, d’autre part, nous devons, en tant que responsables politiques, redoubler d’humilité et de sens des responsabilités. L’accord de Nouméa prévoit qu’en cas de réponse négative à la question posée, « les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée ». C’est le processus qu’a engagé le Gouvernement ces deux dernières années, avec des fortunes diverses. Aujourd’hui, le dialogue entre l’État et les indépendantistes est – hélas ! – quasiment rompu : l’Union calédonienne, principale formation politique du FLNKS, a décidé de ne plus participer

de loi organique que nous examinons aujourd’hui est un texte assez simple, « anodin » comme l’a dit le rapporteur, qui prévoit de reporter les élections provinciales à une date non précisée,

Le second texte, de nature constitutionnelle, concerne le corps électoral spécial et son dégel. Ce sujet occupe une place centrale dans les discussions en cours, puisque c’est ce corps électoral spécial, issu de l’accord de Nouméa et gelé depuis 2007, qui sera amené à participer aux prochaines élections provinciales.

Dans son avis du 7 décembre 2023, le Conseil d’État a rappelé qu’il était nécessaire de revenir à un corps électoral provincial glissant, les dispositions actuelles comportant « des dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage » qu’il convient de modifier afin « d’en corriger le caractère excessif résultant de l’écoulement du temps Le dépôt d’un texte constitutionnel ne traitant que de la question du dégel du corps électoral spécial, que le Sénat devrait examiner à la fin du mois de mars, est loin de faire l’unanimité, contrairement au report que nous examinons aujourd’hui. Il s’agit d’une solution « partielle et unilatérale », qui, au lieu d’aiguillonner le dialogue entre les différentes parties prenantes, comme vous l’aviez évoqué en commission, monsieur le ministre, va au contraire contribuer à aggraver les tensions. Il nous semble en conséquence opportun de nous interroger sur la temporalité envisagée pour l’examen de ce texte, d’autant plus que le report des élections proposé par le Gouvernement doit donner aux différentes parties plus de temps pour parvenir à un accord sous l’égide de l’État, à un consensus s’inscrivant dans un cadre républicain et démocratique. Le cadre républicain, c’est l’accord de Nouméa qui a été constitutionnalisé et approuvé par 72 % des Calédoniens. Il doit constituer le plancher de ce nouveau consensus. Le cadre démocratique, c’est le résultat des consultations référendaires, l’expression de la souveraineté du peuple calédonien sur son avenir, qui doit en constituer le plafond. La mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle Calédonie avait d’ailleurs souhaité que les différents sujets institutionnels ne soient pas traités de manière isolée, en silos, et avait marqué sa nette préférence pour un accord global. Cette position est également celle du Conseil d’État, qui considère que la recherche du consensus, poursuivie depuis vingt par les gouvernements successifs constitue une donnée fondamentale de l’élaboration de l’organisation politique qui prendra la suite de celle issue de l’accord de Nouméa. Les heurts qui se sont déroulés la semaine dernière ont constitué un exemple, si besoin en était, du contexte particulièrement préoccupant sur l’île. votera évidemment le projet de loi organique qui nous est présenté aujourd’hui. Pour autant, nous appelons de nos vœux, monsieur le ministre, une nouvelle initiative. Nous savons que vous êtes déjà beaucoup engagé sur ce

demeure traversée par de profondes inégalités dans tous les domaines. Ces inégalités sont le miroir de l’histoire coloniale. On constate ainsi un décrochage scolaire beaucoup plus important parmi les élèves dont la langue maternelle n’est pas le français, mais aussi des inégalités en termes de revenus ou d’occupation des postes à responsabilité dans l’économie – et j’en passe. Ces problèmes ne peuvent évidemment pas être résolus dans le cadre du statut actuel, qui a toujours été conçu, nous le savons, comme transitoire. Vingt cinq ans après la signature de l’accord de Nouméa, il est temps que ce statut évolue. C’est pourquoi les négociations en cours réunissant tous les acteurs locaux et l’État sont essentielles. Dans l’esprit de la démocratie consociative, qui a permis de bâtir des ponts sur les fractures profondes, ces échanges doivent permettre un accord de long terme sur un nouveau statut

même été élue dans le cadre d’un scrutin reporté d’un an à cause de la pandémie du covid 19. Cette décision a fait mal au processus en cours. À l’époque, le ministre des outre mer, Sébastien Lecornu, avait déclaré : « En démocratie, les élections se tiennent à l’heure.

mais cette évolution doit impérativement être négociée avec tous les acteurs. La procédure actuelle pourrait éventuellement être envisageable si le contenu de la réforme était consensuel, mais ce n’est manifestement pas encore le cas. La réforme du corps électoral proposée par le Gouvernement ne peut pas aboutir, tout du moins

de toutes les questions qui en découlent devraient intervenir à la suite d’un accord politique, et non en amont. La parole

le temps de modifier la Constitution pour ouvrir plus largement le corps électoral et d’organiser le scrutin qui doit normalement se tenir en mai 2024. Le Gouvernement, en facilitant l’intégration des nouveaux arrivants en prévoyant une durée de résidence de dix ans, cherche à légitimer une nouvelle forme de colonisation de peuplement en organisant une noyade démographique du peuple originel. C’est totalement contraire aux résolutions des Nations unies, qui recommandent aux « puissances administrantes » de « veiller à ce que l’exercice à l’autodétermination ne soit pas entravé par des modifications de la composition démographique dues à l’immigration ou au déplacement de populations dans les territoires qu’elles administrent Dorénavant, le gouvernement français décide seul, au nom de la démocratie, qui sera citoyen calédonien et met ainsi fin aux équilibres ardemment négociés entre partenaires calédoniens. Souvenons nous que l’ouverture du droit à l’autodétermination aux communautés arrivées par la colonisation est le fruit de l’accord de Nainville les Roches en juillet 1983. Souvenons nous que la citoyenneté calédonienne a été un enjeu essentiel de l’accord de Nouméa. Aujourd’hui, avec ce projet de loi, la question de la citoyenneté calédonienne est définitivement et unilatéralement préemptée par l’État. Le Gouvernement veut ainsi revenir sur la réforme constitutionnelle de 2007 engagée par Jacques Chirac qui, lui, nous avait compris et dont je salue la mémoire. Lors

cette méthode semble révolue. Sous prétexte d’encouragement au dialogue, le Gouvernement accélère la cadence et veut prendre de vitesse l’opinion française et le peuple kanak par la même occasion. La justification maladroite du projet de loi montre que l’objectif du report n’est pas de faciliter les discussions. Ce changement brutal de méthode suscite de très vives inquiétudes.

De même, ils ont dénoncé la légèreté avec laquelle sont traités des éléments fondamentaux de l’accord de Nouméa, qui n’appartiennent qu’aux discussions entre partenaires locaux. La volonté de l’État de contraindre les partenaires indépendantistes à conclure absolument un accord global avant le 1 juillet ignore le temps du palabre.

Nous déplorons que cet esprit, qui a contribué à déployer le vivre ensemble, n’anime plus nos interlocuteurs actuels. Le Gouvernement a choisi son camp et remet en cause le corps électoral, qui est l’essence même de ce processus novateur et inédit de décolonisation.

considère que les circonstances locales perdurent au regard des droits de l’Homme aussi longtemps que notre pays reste sur la voie de la décolonisation. Les élections provinciales pourraient donc, sans ambiguïté,

de la troisième consultation n’aurait il pas été tout aussi exceptionnel et transitoire ? Un poids, deux mesures ! Et nous sommes de nouveau devant ce dilemme : si la démocratie se révèle être un obstacle à la décolonisation, laquelle de ces deux notions devient prioritaire ? Il n’y a pas de réponse prédéfinie. La réponse, une fois de plus, devrait être donnée par l’histoire. Chez nous, le temps du palabre est plus profitable que la témérité. Le Président du Sénat l’a lui même rappelé, lors de notre première rencontre : le temps du palabre est un temps de sagesse.

les affrontements identitaires du milieu des années 1980 entre Kanaks et Caldoches sont encore présents dans nos esprits. Les accords de Matignon, en 1988, puis ceux de Nouméa ont permis de ramener la paix sur le territoire et d’ouvrir un nouveau chapitre institutionnel et politique. Nous sommes amenés aujourd’hui à nous réinterroger sur la structure du corps électoral de l’archipel, qui a forcément évolué depuis cette période. Dès lors, nous considérons que ce projet de loi organique satisfait les exigences des parties engagées dans le processus d’accession à la pleine souveraineté prévu par l’accord de Nouméa et étalé sur vingt ans. Nos débats, portant strictement sur l’examen d’un texte qui reporte l’échéance d’élections, ne peuvent se mettre en retrait d’un contexte plus général relatif au dégel du corps électoral. Le principe de restriction qui valait jusqu’alors était justifié par la reconnaissance de la citoyenneté calédonienne en complémentarité de celle de la nationalité française. Désuet, il constitue aujourd’hui une dérogation, si ce n’est une atteinte au principe d’universalité du suffrage fixé par l’article 3 de notre Constitution. en ce début d’année, les dispositions actuelles continueraient d’exclure du vote un certain nombre d’électeurs pourtant nés et résidant depuis plusieurs décennies sur la Grande Terre.

Le RDSE tient à saluer les efforts de toutes les parties pour faire accéder l’île et ses habitants à une plus grande sérénité institutionnelle, sociale et économique – sérénité évidemment sous tendue par nos discussions. En effet, ces textes ouvriront une ardente bataille politique dans les assemblées locales et au congrès autour du processus d’autodétermination, sur la base du travail tripartite achevé en septembre dernier. Ces projets de loi nous donnent une échéance, un horizon, pour nous laisser le temps de réfléchir à cette question : jusqu’où adapter le modèle républicain pour que la Nouvelle Calédonie demeure française, si elle le demeure ? Observons ici que bon nombre de femmes et d’hommes de par le monde aspirent à accéder à la nationalité française, et qu’il est surprenant que d’autres s’interrogent sur celle ci ou rêvent de s’en libérer Le Gouvernement doit être en mesure de se saisir des travaux du Sénat, notamment des conclusions de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle Calédonie. Nous serons particulièrement vigilants sur les points d’achoppements des deux parties. Les trois référendums passés ont laissé des plaies encore béantes et les clivages se sont considérablement accentués. Dans ce contexte, monsieur le ministre, il est tout à fait légitime que le Sénat vous demande des garanties sur la sérénité des discussions en cours. L’État doit être impartial et transparent, l’État doit être loyal, l’État doit être intransigeant, pour préserver la sûreté de tous les citoyens calédoniens. Les auditions conduites par nos collègues l’ont montré

Cela m’interpelle. Certes, les nombreux déplacements de délégations métropolitaines vers l’archipel, ces derniers mois, vont dans le bon sens. Mais comment ne pas prendre en compte cet inquiétant facteur dans l’équation géopolitique de l’Indo Pacifique, complexifiée par la stratégie agressive de la République populaire de Chine ? Le désir d’indépendance ne doit pas occulter l’équilibre très précaire qui règne dans la région. L’avenir de l’archipel ne peut s’organiser sans mettre en place une coopération renforcée dans les secteurs économiques, énergétiques et sociaux, déjà en souffrance. Enfin, le Sénat y tient beaucoup : l’avenir doit s’écrire avec tous les acteurs et respecter le processus démocratique exigeant, à la hauteur de la devise du Caillou qui a été rappelée par notre collègue Hervé Marseille : terre de parole, terre de partage. Le groupe du Rassemblement Démocratique et Social

le texte qui nous est soumis aujourd’hui prévoit le report des élections provinciales de Nouvelle Calédonie du mois de mai à une date non précisée, mais qui ne pourra pas excéder le 15 décembre 2024. Il prévoit également le prolongement, par voie de conséquence, du mandat en cours des membres du congrès et des assemblées de province élus le 12 mai 2019. Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, les élections peuvent être reportées et le mandat des élus concernés prolongé, dès lors que la mesure est justifiée par la poursuite d’un intérêt général et qu’elle n’est pas disproportionnée. Le Conseil d’État a estimé, dans ses avis du 7 décembre 2023

En effet, le corps électoral pour ces élections est gelé depuis la réforme constitutionnelle du 23 février 2007. Il en résulte qu’en 2022 près de 20 % des électeurs, soit 41 679 personnes, étaient inscrits inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle Calédonie sans pour autant être inscrits sur la liste électorale spéciale pour les élections provinciales. Or les provinces exercent de larges compétences. Organiser un scrutin sur cette base électorale restreinte pourrait entraîner des conséquences en droit électoral que personne ne souhaite. Il revient donc aux forces politiques calédoniennes de s’entendre pour déterminer la composition, dont on connaît l’importance et la spécificité pour ce territoire, du corps électoral appelé à voter pour les prochaines élections provinciales.

Il vous appartenait néanmoins, monsieur le ministre, de parer à l’éventualité d’un échec des discussions. Aussi avez vous déposé, le 29 janvier dernier, un projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral pour les élections provinciales et l’ouvrant aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle Calédonie, sont nés sur ce territoire ou y sont domiciliés depuis au Cette révision constitutionnelle entrerait en vigueur le 1 juillet 2024, après adoption par le Parlement réuni en Congrès, sauf si un accord politique et institutionnel était conclu entre les partenaires avant cette date – ce qui reste, bien évidemment, l’objectif premier du Gouvernement. L’atmosphère dans laquelle s’est déroulé votre récent déplacement dans l’archipel ne doit pas faire oublier l’attention particulière que le Gouvernement a portée aux positions exprimées par les membres du congrès de la Nouvelle Calédonie, y compris y compris ceux qui ont exprimé des réticences vis à vis de toute révision du corps électoral, pour construire une solution pacifiée. Pour conclure,

Elle nous l’a démontré à plusieurs reprises : en 1988 avec les accords de Matignon, puis en 1998 avec ceux de Nouméa. Elle nous l’a montré alors même que s’étaient produits des conflits si lourds et si tragiques. Je suis certain qu’elle saura dépasser les clivages, cette fois encore, pour parvenir à un accord qui satisfasse l’ensemble des forces en présence. Comparaison n’est pas raison, mais je sais ce que c’est que d’appartenir à un territoire singulier. C’est pourquoi je veux assurer les Calédoniens

et ce pour plusieurs raisons. D’abord, le Gouvernement a fait le choix de lier le sujet du report des élections au projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. Or ce dernier sujet, le corps électoral, est la clé de voûte des accords trouvés jusqu’ici. Sans cet élément majeur dans la construction de la paix en Nouvelle Calédonie, c’est un compromis qui risque de s’effondrer – et je pèse mes mots.

sujet dépasse même les 270 000 habitants de l’île, car la méthode utilisée par le Gouvernement est contre productive. Les accords de Matignon, sous le Gouvernement de Michel Rocard, ou encore les accords de Nouméa, sous Lionel Jospin, ont pu être trouvés grâce à une logique de consensus, grâce à un credo : la discussion, encore et toujours, comme pilier de la résolution des conflits.

C’est donc une rupture totale de méthode à laquelle nous faisons face ; cela ne correspond ni à l’histoire de ce territoire ni à l’esprit qui a conduit jusqu’ici aux solutions de paix. Le sujet qui nous anime est celui de la décolonisation et son corollaire : quelle forme d’autodétermination ? Plus largement, c’est aussi la question du droit à l’émancipation qui nous est posée aujourd’hui. Ce ne sont pas là de vains mots, surtout pour la Nouvelle Calédonie qui a une histoire complexe, parfois troublée, avec des drames faits de larmes et de sang.

et de la plus grande neutralité, seules garantes de son rôle central et de la tenue de débats internes sereins. En imposant une solution, en imposant des délais courts, le Gouvernement ne respecte plus ces préceptes et opère un changement de paradigme que j’estime dangereux. Quand la réflexion est contrainte, il ne reste souvent plus que l’émotion, qui est rarement bonne conseillère. Les accords de Matignon comme de Nouméa

Les choix opérés depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron démontrent une partialité délétère. Ainsi, en 2021, comme cela a été rappelé plusieurs fois déjà,

à constater l’impossibilité de tenir des élections et donc à être favorables au report. Il faut donner du temps au temps et, en Nouvelle Calédonie, mes chers collègues, ce temps est nécessairement très long. La parole est

lier leur destin à celui de la République. Mais, dans notre assemblée, acquise à la décentralisation, nous savons qu’on ne pilote pas une collectivité à 17 000 kilomètres de distance. Les sénateurs du groupe Les Républicains soutiendront ce projet de loi organique reportant au plus tard au 15 décembre 2024 l’élection des membres du congrès et des assemblées de province En effet, ce report s’inscrit dans le cadre plus large des négociations lancées après l’achèvement du processus politique balisé par l’accord de Nouméa et marqué, je le rappelle, par le troisième vote défavorable à l’indépendance du 12 décembre 2021. Depuis cette date, les discussions entre acteurs calédoniens, mais aussi avec l’État, se poursuivent et s’intensifient avec pour objectif d’aboutir à un accord politique global et consensuel. Ces discussions, difficiles, n’ont malheureusement pas encore abouti. Pourtant, leur conclusion positive le gage d’un avenir institutionnel serein pour le Caillou et le maximum doit être fait afin d’en réunir les conditions. Évidemment, le déroulement, en parallèle, d’une campagne électorale, suivie du renouvellement des assemblées provinciales et du congrès, risquerait de parasiter les négociations, d’autant plus que les mécanismes institutionnels sont eux mêmes l’un des points de la discussion. Or, la date de ces élections étant fixée au 12 mai 2024, il n’est pas réaliste d’envisager de conclure dans ce délai. Non seulement l’enchaînement d’un hypothétique accord et du scrutin serait délicat sur le plan pratique, mais un tel empressement serait presque certainement nuisible à la sérénité des travaux. Si nous voulons donner une chance au dialogue, ce report s’impose donc. L’objectif d’intérêt général justifiant de différer la date des élections est indéniable, comme l’ont considéré le Conseil d’État dans ses récents avis ainsi que notre rapporteur, Philippe Bas, fin connaisseur du sujet, dont je salue les conclusions. En outre, la consultation ce projet de loi organique a démontré que le report était largement approuvé par les élus du territoire, puisque les deux tiers d’entre eux se sont exprimés en sa faveur. Quoiqu’il paraisse difficile de dire avec certitude si un accord sera trouvé d’ici décembre, la commission a estimé préférable de s’en tenir, à ce stade, à la date proposée par le Gouvernement, position partagée par les sénateurs du groupe Les Républicains. J’aborderai également la question du corps électoral. Souvenons nous que la création d’un corps électoral spécial était une dérogation d’une telle ampleur au principe d’égalité devant le suffrage qu’elle avait nécessité de modifier la Constitution. Son évolution nécessitera donc une nouvelle

À ce sujet, je tiens d’ailleurs à m’associer au souhait exprimé en commission des lois d’inscrire le futur texte constitutionnel dans le cadre d’un accord global entre les partenaires calédoniens. Un tel compromis est plus indispensable que jamais pour l’avenir de ce territoire qui fait face à d’importants défis économiques et sociaux – l’incertitude institutionnelle ne rend que plus compliqué de les relever. La fragilité de la filière nickel en est une illustration. Pour leur développement, nos collectivités ont certes besoin d’un cadre institutionnel adapté et accepté. Mais cela ne constitue qu’un préalable et non un aboutissement. Pour faire exister le rêve français jusqu’en mer de Corail, nous devons offrir des perspectives à la jeunesse insulaire. Et la prospérité de demain se bâtit aujourd’hui, en faisant travailler ensemble le Gouvernement, le Parlement, les élus et les forces vives de la Nouvelle Calédonie ! La discussion

de préserver l’esprit des accords de Matignon et de Nouméa. Il tend également à formuler une mise en garde. En premier lieu, il rappelle que la méthode de discussion entre les partenaires, adaptée à chaque fois aux circonstances nouvelles, apparaît comme une donnée structurante, un cadre intangible intangible et contraignant, qui s’impose aujourd’hui à l’action des femmes et des hommes impliqués dans l’évolution institutionnelle de la Nouvelle Calédonie pour définir l’après accord de Nouméa. Le temps de la discussion et du compromis constitue une variable déterminante dans l’histoire récente de ce territoire. Cette méthode a fait ses preuves, en rétablissant et en maintenant la paix civile, en faisant en faisant fonctionner des institutions spécifiques, en engageant le rééquilibrage en matière de développement économique et de formation et en permettant d’insérer la Nouvelle Calédonie dans son environnement régional. Il s’agit également d’une méthode qui témoigne de la confiance accordée aux responsables politiques de la Nouvelle Calédonie. Ceux ci font preuve d’un grand sens des responsabilités et d’une profonde maturité politique, qui ont toujours permis de surmonter les moments de doute ou de découragement. Aujourd’hui, l’option retenue par le Gouvernement est à l’opposé de cette démarche constructive et pragmatique, qui s’appuie sur la réalité de la destinée de la Nouvelle Calédonie et qui rejette toute décision imposée unilatéralement sans profiter à personne. Si le Gouvernement persiste dans cette voie inappropriée en maintenant le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral déposé dans le prolongement du présent projet de loi organique, il engage sa responsabilité au premier chef. À chaque fois qu’il donne le sentiment d’être sorti de sa neutralité, il laisse la place aux tensions, qui risquent de s’aggraver, comme on a pu le constater à Nouméa lors du dernier déplacement du ministre de l’intérieur en Nouvelle Calédonie. Nous appelons une fois de plus à de nouvelles initiatives pour retrouver la voie du consensus et de la conclusion d’un accord global.

et je dois vous dire qu’elle en partage la bienveillance. En effet, la commission des lois tout entière souscrit

aux gouvernements qui se sont succédé depuis les accords de Matignon et de Nouméa que de considérer qu’ils n’ont pas tous été guidés par la recherche du consensus,

Je rappelle que la consultation de décembre 2021 a été demandée par les indépendantistes en avril 2021 et que sa date a été fixée après avis favorable du congrès. Parvenir à un accord global a toujours été et demeure l’objectif prioritaire du Gouvernement. Ce dernier a multiplié les échanges bilatéraux avec chacun des deux camps, à Nouméa comme à Paris. Conformément à la demande du FLNKS, un bilan d’ensemble de l’accord de Nouméa et un audit de la décolonisation ont été menés, afin que ces documents servent de base aux discussions sur l’avenir institutionnel

J’y ai passé cinq jours et j’ai fait un certain nombre d’annonces en matière d’immobilier judiciaire et de renforcement des ressources humaines et dans le domaine pénitentiaire. Je ne crois pas que l’État soit d’une quelconque manière défaillant pour tenter de faire émerger une solution équilibrée, consensuelle et durable. Le Président de la République a exprimé cette volonté avec force lors de son voyage officiel à Nouméa en juillet dernier, en invitant l’ensemble des Calédoniens à définir eux mêmes le chemin de l’avenir,

Néanmoins, il n’est nullement utile de l’inscrire dans le corps même de ce projet de loi, qui vise uniquement à reporter la date des élections provinciales. C’est pour cette raison que je voterai contre cet amendement et que j’invite mes collègues de la majorité sénatoriale à s’y opposer

Le rapporteur, qui s’est rendu en Nouvelle Calédonie avec le président de la commission, François Noël Buffet, et Jean Pierre Sueur dans le cadre d’une mission de la commission des lois, a estimé que la conclusion d’un accord global constituait une condition déterminante pour l’approbation finale d’un accord par le Parlement une révision constitutionnelle et l’adoption d’un projet de loi organique portant un statut renouvelé de la Nouvelle Calédonie. Compte tenu de ces considérations, notre groupe reprend à son compte l’interrogation que le rapporteur a exprimée au ministre de l’intérieur à l’occasion de son audition devant la commission des lois. mesure où les discussions entre les formations indépendantistes et non indépendantistes ont débuté bien avant la présentation du projet de loi constitutionnelle, ne serait il pas plus avisé de leur laisser davantage de temps, ne puissent pas nous soupçonner d’exercer une pression sur elles en adoptant un texte comportant une solution à la fois unilatérale et partielle ? Si nous estimons que le report des élections

Retarder des élections, c’est forcément différer le fonctionnement normal de la vie démocratique. Je comprends que le Gouvernement

Le Gouvernement travaille sans relâche depuis plus de deux ans pour tenter de faire émerger un accord global qui poserait les bases d’un nouveau statut. La question du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province constitue l’un des points de crispation les plus forts en Nouvelle Calédonie. d’un consensus dans le cadre d’un accord global sur ce point aurait été évidemment la meilleure des options. De fait, il a fallu attendre que le Gouvernement dépose ces deux projets de loi pour que les négociations progressent.

Le Gouvernement a clairement indiqué qu’interdire à des citoyens qui sont présents sur le territoire depuis vingt cinq ans, ou qui y sont nés, de participer à la vie démocratique locale n’était plus conforme aux exigences d’un État démocratique ni aux engagements internationaux de la France. Il a été tout aussi clair sur le fait que, faute d’un accord global entre les partenaires avant le 31 décembre 2023, il proposerait au Parlement un dégel du corps électoral sur la base médiane d’un temps de résidence

qui est aussi celle du Gouvernement, de ne rien vouloir brusquer. Je tiens à vous rassurer. Le projet de loi constitutionnelle prévoit, par un mécanisme à double détente, que le Gouvernement puisse décider d’un nouveau report des élections dans l’hypothèse où un accord serait conclu entre l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle et la nouvelle date du scrutin. Votre préoccupation me semble donc ainsi prise en compte. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Le territoire traverse une crise économique d’une ampleur sans précédent, qui impose des décisions fortes. Celles ci doivent être prises le plus rapidement possible, par des assemblées renouvelées par le suffrage des Calédoniens. Vous évoquez également l’avis du Conseil d’État de décembre 2023. Au regard des exigences constitutionnelles, un report à novembre 2025 est effectivement possible techniquement, mais il n’est souhaitable ni politiquement ni démocratiquement.

Le report des élections ne doit se comprendre qu’au regard de la révision constitutionnelle qui permettra de rétablir l’égalité devant le suffrage : les modalités de ce dernier ne satisfont plus aux exigences constitutionnelles et conventionnelles qui nous engagent.

nous avons tous pris la mesure de l’importance que ce texte revêt au regard de la situation politique de cet archipel français du Pacifique. Ce report est en effet indispensable et nous ne pouvons le comprendre qu’à la lumière de la révision constitutionnelle qui interviendra dans les prochaines semaines

modifier les dispositions qui instaurent une injustice pour des milliers de Calédoniens de cœur ou de naissance qui, aujourd’hui, ne sont pas autorisés à voter aux élections provinciales.

Songez, mes chers collègues, qu’en Nouvelle Calédonie des milliers de citoyens français, qui y sont nés, qui ont aujourd’hui entre 18 et 25 ans et qui y ont vécu toute leur jeunesse, se voient refuser le droit de vote aux élections provinciales, car leurs parents se sont installés sur le impossible que les prochaines élections provinciales aient lieu dans deux mois dans ces conditions. Différons les ! Tel est l’objectif de ce projet de loi. Révisons la Constitution, dégelons le corps électoral provincial, intégrons les électeurs qui répondent aux nouveaux critères de définition d’un corps électoral évoluant de manière glissante dans le temps. C’est seulement après que nous pourrons organiser sans délai les élections provinciales. C’est pourquoi je voterai en faveur de ce projet de loi organique et je vous invite, mes chers collègues, à en faire de même le plus largement possible

La date de décembre me semble tout à fait raisonnable. Comme cela a été dit par certains de mes collègues, la situation économique et sociale de la Nouvelle Calédonie ne nous permet pas de perdre plus de temps

commission, l’ensemble du projet de loi organique portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle Calédonie. En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

La séance est suspendue. La séance est reprise. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement

madame la rapporteure pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est un honneur pour moi de venir devant vous, pour la première fois, présenter et défendre un texte du Gouvernement. En tant qu’ancien parlementaire et ancien président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, je suis particulièrement sensible à l’engagement et à l’implication des parlementaires, notamment des membres de cette assemblée, sur la question cœur battant de la démocratie et des territoires. Ils sont au centre de la construction de la loi. J’en suis intimement et profondément convaincu. Je tiens à remercier les membres des deux commissions saisies, qui ont adopté ce texte tout en l’enrichissant nettement.

à améliorer et à renforcer le traitement de l’habitat dégradé dans notre pays. Je veux tout particulièrement saluer l’engagement et l’implication de Mme la présidente Dominique Estrosi Sassone et de Mme la rapporteure Amel Gacquerre, avec qui nous avons eu des échanges constructifs, malgré des délais contraints : voilà qui présage, j’en forme le vœu, d’échanges aboutis sur d’autres sujets à l’avenir. Je souhaite également remercier l’ensemble des sénateurs, qui ont manifesté leur intérêt prononcé sur ce texte et, de manière générale, leur volonté de travailler avec le Gouvernement et mes équipes pour répondre à la crise du logement.

Conformément à la volonté exprimée par le Président de la République de prendre des mesures d’exception pour produire plus rapidement des logements, le Premier ministre a demandé à son gouvernement d’accélérer et de simplifier toutes les procédures en la matière, afin de créer un choc d’offre dans le secteur. C’est un point sur lequel nous commençons à agir dès ce premier texte, comme en témoigne l’article 14 qui comporte des leviers, auxquels je suis particulièrement attaché, pour accélérer la production de logements dans les territoires où les besoins sont les plus forts.

ce programme important permettra, dans les trois prochaines années, d’accélérer la construction de 30 000 logements dans vingt deux territoires où les enjeux sont particulièrement importants.

à l’avenir, aux collectivités, aux opérateurs et à l’État de traiter plus rapidement et avec plus d’agilité les situations de dégradation financière et bâtie qui caractérisent notre parc d’habitat et qui ont des effets sur la vie de nos concitoyens. Il est tout simplement intolérable que des personnes continuent de vivre aujourd’hui, dans notre pays, dans des conditions d’habitat dégradé, indécent ou indigne. Près de 1,5 million de logements sont dégradés : ce sont autant de foyers et de familles qui connaissent des situations de vie inacceptables. Avec ce texte, nous nous attaquons directement à ce problème, en aidant les copropriétés à emprunter les sommes nécessaires pour faire les travaux de rénovation, en renforçant les outils à la disposition des élus et des opérateurs pour mener de grands projets de réhabilitation et en augmentant les sanctions contre ceux qui mettent à profit la dégradation de l’habitat. C’est la continuation d’un travail que nous avons entamé dès 2017. Mes prédécesseurs en ont fait une priorité de leur action : Julien Denormandie a ainsi lancé, dès 2018, le plan Initiative Copropriétés (PIC) pour s’attaquer aux cas des grandes copropriétés en difficulté.

Mathieu Hanotin, maire socialiste de Saint Denis, et Michèle Lutz, maire Les Républicains de Mulhouse, pour explorer les moyens d’améliorer la prise en charge de ces situations difficiles. Leurs travaux ont permis à mon prédécesseur, Patrice Vergriete, d’élaborer le texte qui vous est soumis, et qui a pour objet de mettre à la disposition des collectivités des outils pour enrayer et traiter la dégradation de l’habitat. Nos efforts ont porté sur deux axes majeurs, qui se retrouvent dans les deux chapitres de ce projet de loi. Il faut, d’une part, que nous anticipions mieux les situations de dégradation, qui mettent plusieurs années à s’installer et peuvent donc faire l’objet d’un traitement plus en amont. Pour cela, il est indispensable d’avoir une vision prospective afin de mieux prévenir l’émergence de dynamiques de fragilisation et d’intervenir plus tôt grâce au professionnalisme et à la mobilisation de tous les acteurs concernés. Dans cette optique, le projet de loi crée notamment, à l’article 3, une nouvelle procédure d’expropriation qui permettra d’intervenir en amont du cycle de dégradation. Cette faculté, à la main des collectivités et de l’État, concernera les immeubles qui sont frappés par un arrêté de police, mais qui ne sont pas encore, pour autant, dans une situation de dégradation irrémédiable.

Je tiens à le souligner, c’est une innovation majeure, qui a d’ailleurs soulevé un débat avec les banques et les professionnels, débat qui va certainement se poursuivre dans les semaines à venir. Il s’agit d’un outil de simplification bienvenu pour surmonter les blocages et les difficultés inhérentes aux travaux dans les copropriétés. Il fera gagner plusieurs mois dans de dossiers individuels, au profit d’une approche collective et globale. Au fond, ce prêt peut être, je le crois, l’innovation financière qui manque pour massifier la transition écologique dans chaque microdémocratie qu’est une copropriété. Bien sûr, cela ne peut pas se faire de manière floue,

Il importe, d’autre part, de poursuivre la lutte que nous avons engagée dès 2017 contre les marchands de sommeil et de renforcer les sanctions à leur encontre. Les marchands de sommeil sont des délinquants qui tirent une rente de la vulnérabilité des personnes. Sur l’initiative du député Lionel Royer Perreaut, corapporteur du texte et élu d’un territoire très marqué par ce phénomène, l’Assemblée nationale a ajouté des dispositions importantes en la matière. Je veux remercier ici les sénateurs d’avoir largement repris et enrichi ces mesures, qui sont cruciales pour notre dignité collective. De manière générale, je tiens à saluer l’esprit de consensus qui a guidé les travaux sur ce texte dans les deux assemblées. Cela montre à quel point la conscience de ces difficultés traverse les partis et dépasse les positionnements politiques. Par ailleurs, il faut que nous traitions plus rapidement les dégradations les plus marquées avant qu’elles n’aboutissent à des situations d’indignité insupportables et irrémédiables. Nous devons éviter au maximum d’arriver à la situation dans laquelle démolir pour reconstruire est plus intéressant financièrement que rénover et réparer. Pour cela, nous souhaitons accélérer l’ensemble des procédures de recyclage et de transformation des copropriétés, qui prennent aujourd’hui trop de temps. En effet, aujourd’hui, tous les acteurs en conviennent, les délais des opérations de réhabilitation sont beaucoup trop importants. Il faut parfois jusqu’à quinze ou vingt ans pour mener à bien un projet, ce qui provoque l’incompréhension des habitants et des élus, leur lassitude, et même la souffrance des propriétaires et des occupants qui se retrouvent dans des situations provisoires à durée indéterminée. Plusieurs mesures de ce texte permettront d’accélérer de façon décisive les opérations de transformation. C’était la volonté du Président de la République, qui l’avait dit très clairement lors de son déplacement à Marseille à la fin du mois de juin dernier. Le déroulement des opérations de traitement de la dégradation sera fluidifié par une meilleure capacité à répondre aux besoins de relogement inévitables qui en découlent. Ainsi, le maire pourra autoriser l’implantation, sans permis de construire, de logements temporaires pour reloger les personnes délogées par les chantiers. Tel est l’objet de l’article 7 . Le maire pourra aussi faire réaliser, aux frais du propriétaire, la remise en état de biens lorsque des travaux ont été menés de façon irrégulière – c’est l’article 3 . Les articles 11 et 12 permettront quant à eux d’accélérer et de sécuriser les expropriations menées dans le cadre de la législation dite Vivien, qui est engagée lorsque des bâtiments sont atteints d’une dégradation irrémédiable. Toutes ces mesures sont autant d’avancées opérationnelles souhaitées, parfois de très longue date, par les professionnels et les élus des territoires concernés. C’est la raison pour laquelle je souhaite vivement, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous puissions travailler ensemble pour enrichir ce projet de loi et en faire un levier d’accélération, de simplification et de rénovation encore plus performant. Avec ce texte, donnons nous les moyens de répondre à la crise du logement de manière pragmatique, opérationnelle et transpartisane, en nous attaquant aux problématiques des copropriétés dégradées, de la sécurité et de la qualité des logements. Enfin, je forme le vœu que ce texte ne soit que la première étape d’une longue série de travaux partagés pour répondre ensemble aux défis du logement. La parole

le projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, que nous examinons à partir d’aujourd’hui, est un texte certes technique, mais qui ne doit pas faire oublier la réalité des copropriétés fragilisées ou dégradées de nos territoires. Une réalité qui conduit les maires à nous demander de leur redonner le pouvoir d’agir. Vous le savez,

de centres villes ou centres bourgs anciens. Or les maires sont trop souvent démunis face à la complexité des procédures à mettre en œuvre. Surtout, la longueur de ces procédures laisse prospérer les marchands de sommeil et se développer l’habitat indigne, jusqu’à aboutir parfois à de tragiques effondrements d’immeubles, comme ceux de la rue d’Aubagne, à Marseille. Pour ma part, j’ai une idée simple : il faut simplifier pour accélérer. Il faut pouvoir aboutir en un mandat municipal et non en deux, trois voire quatre

Sur le premier volet, nous avons souhaité faciliter le travail de tous les maires, y compris dans les petites communes. Tout d’abord, nous avons intégré dans les missions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) le conseil et le soutien aux collectivités territoriales en faveur de la rénovation de l’habitat dégradé, tout particulièrement lorsque celles ci n’ont pas de services dédiés suffisants. Nous avons aussi souhaité donner davantage d’outils aux maires pour prévenir la dégradation de l’habitat. Prolongeant une mesure introduite à l’Assemblée nationale, nous leur avons ainsi donné le pouvoir de faire réaliser d’office un diagnostic structurel des immeubles dans les zones d’habitat dégradé aux frais des propriétaires. La commission des affaires économiques a aussi eu à cœur de faciliter les procédures. Notre idée force est de permettre la mobilisation des dispositifs disponibles plus en amont, avant que la démolition ne devienne inéluctable. restauration immobilière (ORI) ont été retravaillées en ce sens, et le texte crée une nouvelle procédure d’expropriation pour les immeubles dégradés à titre remédiable. Cette mesure était très attendue par les maires, pour qui la procédure d’expropriation Vivien, prévue pour les immeubles indignes à titre irrémédiable, est souvent trop difficile à mettre en œuvre. Le texte étend aussi la possibilité pour les collectivités de recourir à des concessions d’aménagement dans le cadre d’opérations de résorption de l’habitat indigne, y compris ponctuelles, ponctuelles, ce qui est très précieux pour les communes manquant d’ingénierie. Toutes ces évolutions ont reçu un soutien unanime, tant des élus locaux que des aménageurs et autres parties prenantes. La commission des affaires économiques s’est efforcée d’élargir ou de préciser le champ d’utilisation de ces dispositifs afin de faciliter leur mise en œuvre pour les petites copropriétés dégradées de nos centres bourgs ou de nos centres villes anciens, pour lesquelles il existe peu ou pas d’outils d’aménagement spécifiques. Nous avons ainsi élargi le champ de la concession d’aménagement aux immeubles frappés d’arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et aux îlots

La commission des affaires économiques a aussi adopté plusieurs amendements visant à sécuriser les procédures d’expropriation, notamment des immeubles dégradés à titre remédiable, en précisant les les modalités de réduction de l’indemnisation pour tenir compte de l’état de dégradation du bien. Nous souhaitons également assurer une meilleure protection des occupants. Elle a aussi prolongé une disposition introduite par l’Assemblée nationale permettant le relogement d’occupants évincés dans le cadre d’actions d’actions de résorption de l’habitat dégradé dans des constructions temporaires. Nous sommes allés avec pragmatisme au bout de cette logique en supprimant l’échéance des cinq ans. Dans le même temps, nous avons sécurisé le dispositif, à la fois pour les occupants délogés et pour les maires des communes concernées. Je rappelle que plus de 90 % des maires ayant répondu à la consultation en ligne lancée par le Sénat ont soulevé les difficultés posées par le relogement des occupants. C’est un vrai problème, un vrai frein pour le lancement de projets de rénovation de l’habitat dégradé. Si nous voulons accélérer la lutte contre l’habitat indigne, ne nous privons pas de solutions pragmatiques et efficaces. Toujours dans le souci de donner aux maires les moyens d’agir, la commission a introduit dans ce texte la possibilité de mettre gratuitement à leur disposition les immeubles confisqués aux marchands de sommeil pour réaliser des logements.

Nous soutenons pleinement la création d’un nouveau prêt global et collectif aux copropriétés, mais nous sommes convaincus que, pour qu’il soit un succès, il faut que les banques et les organismes de caution puissent s’y engager sans réserve. Pour cela, il faut que la copropriété ne soit pas une boîte noire et que les prêteurs et les cautions puissent respecter leur obligation de « prêt responsable ». Ils doivent pouvoir s’assurer que ce nouveau prêt ne contribuera pas au surendettement des copropriétaires fragiles. Nous sommes tout autant convaincus qu’une contre garantie publique est nécessaire, mais nous ne pouvons pas signer un chèque en blanc au Gouvernement sur un nouveau dispositif sans financement.

C’est une demande forte des maires, confrontés parfois à des syndics ou à des administrateurs provisoires qui ne disposent pas de l’expérience nécessaire pour faire face aux difficultés rencontrées. Nous avons voulu que cette loi permette de constituer dans un premier temps un vivier de syndics volontaires et compétents pouvant prévenir le redressement ou l’accompagner. Il nous faudra faire le bilan de ce dispositif dans quelque temps avant d’aller plus loin. autant, il nous est apparu contraire à la volonté d’efficacité et de simplification qui anime ce texte qu’une forme de « syndic » conduise à une réglementation exagérément alourdie, soupçonneuse, des rapports avec les copropriétaires. la commission des affaires économiques a également souhaité renforcer le volet portant sur la lutte contre les marchands de sommeil, initialement introduit par l’Assemblée nationale. Nous avons ainsi approuvé l’augmentation des peines souhaitées par les députés et je dois dire, monsieur le ministre, que c’est une surprise pour nous d’être en désaccord sur ce point avec l’ancien président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale Nous avons néanmoins réécrit et précisé juridiquement plusieurs mesures importantes, notamment le passage de dix à quinze ans de l’interdiction d’acquérir un bien immobilier encourue par les marchands de sommeil ou encore la possibilité de réprimer le refus d’un bail écrit ou de la remise d’une quittance en cas de paiement en espèces. Il est en effet bien souvent difficile de faire condamner les marchands de sommeil, et les maires nous ont dit que cette nouvelle disposition allait les aider très concrètement Pour lutter contre les marchands de sommeil, nous avons aussi facilité la mise en œuvre des permis de louer et de diviser, outils plébiscités par les maires, et nous avons introduit à titre expérimental la possibilité de déroger en mieux aux règles de droit commun en matière de surfaces et volumes et volumes minimaux de certains logements dans les zones d’habitat dégradé, et ce afin de lutter contre les subdivisions sauvages d’appartements ou de pavillons.

ans presque jour pour jour après l’appel de l’abbé Pierre, l’urgence à agir en faveur d’un habitat digne pour tous reste, malheureusement, pleinement d’actualité. Cette action ne peut ni ne doit laisser de côté les copropriétés : il s’agit d’un enjeu de taille, puisque 40 % des Français y vivent. Or, comme l’ont illustré de trop nombreux exemples assez médiatisés ces dernières années, de nombreuses copropriétés sont dans un état de dégradation avancé, parfois en raison de l’inertie volontaire des marchands de sommeil, ou tout simplement en raison des difficultés financières des copropriétaires ou de blocages en assemblée générale. D’après les chiffres qui nous ont été transmis, 114 000 copropriétés seraient ainsi considérées comme particulièrement fragiles. Dans ce contexte, la commission des lois soutient pleinement l’ambition que porte le projet de loi de moderniser les outils aux mains de l’État, des collectivités territoriales et des opérateurs pour leur permettre d’intervenir le plus en amont possible et ainsi prévenir la dégradation des copropriétés. Parmi les nouveaux outils proposés, je retiendrai notamment la création d’une procédure spéciale d’expropriation pour cause d’utilité publique des bâtiments dont l’état de dégradation ou d’insalubrité est remédiable, sur le modèle de la procédure Vivien, qui permet déjà une expropriation sans enquête publique pour les bâtiments dont l’état de dégradation ou d’insalubrité est irrémédiable. Cette mesure, qui a fait l’unanimité chez toutes les personnes que j’ai auditionnées, permettra ainsi d’intervenir plus facilement tant qu’il est possible de rénover le bâtiment. Je pense également à l’extension des possibilités de scission ou de subdivision judiciaire

garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Nous avons considéré, dans l’ensemble, que le texte atteignait un équilibre satisfaisant entre la facilitation des opérations de rénovation, qui constitue un motif sérieux d’intérêt général, et l’accompagnement des copropriétaires en difficulté, y compris ceux qui seraient récalcitrants. Suivant cette démarche constructive, la commission des lois a émis un avis favorable sur quinze des dix neuf articles dont elle était saisie et a adopté vingt deux amendements, dont dix neuf ont été repris par la commission des affaires économiques et ainsi intégrés au texte qui nous est soumis aujourd’hui. Je tiens à souligner la fluidité et la qualité du travail effectué avec Amel Gacquerre, rapporteure de la commission des affaires économiques. Notre collaboration fut étroite et fructueuse afin de capitaliser sur les compétences de nos deux commissions. Il va donc sans dire que je partage aussi bien les constats que les propos et les préconisations mis en avant à l’instant par notre collègue. Notre seul point de divergence a porté sur le renforcement des sanctions pénales à l’encontre des marchands de sommeil, aux articles 8 et 8 A. La commission des lois s’est en effet prononcée pour la suppression de ces deux articles. Il n’y a, bien évidemment, aucun désaccord sur l’objectif de ces articles, bien au contraire ! La commission des lois s’est d’ailleurs prononcée en faveur des articles qui instaurent des peines complémentaires. Cependant, nous avons relevé que le législateur modifié le quantum des peines applicables à l’encontre des marchands de sommeil voilà à peine un mois, dans le cadre de la loi Immigration du 24 janvier dernier. Il nous a paru nécessaire d’apprécier les effets de ces mesures avant d’en prendre de nouvelles. ailleurs, nous avons estimé qu’augmenter le quantum des peines dans ces proportions posait un problème de cohérence dans l’échelle des peines. Concrètement, cela signifierait que la mise à disposition d’un hébergement indigne serait plus grave que le fait d’être de mauvaise foi dans le respect des obligations de mise de mise en conformité des logements, alors même que l’occupant est une personne vulnérable. Malgré cette divergence d’appréciation, au demeurant minime, la commission des lois soutient pleinement ce texte, qu’elle juge utile autant que nécessaire, et vous invite à l’adopter. La parole

de la rue d’Aubagne. Nous avons notamment travaillé avec Mathieu Hanotin et Michèle Lutz, maires de Saint Denis et de Mulhouse. La commission s’est déplacée à Saint Denis pour mieux comprendre les problèmes concrets. Pour ne donner qu’un seul exemple, nous avons été frappés par le fait que, plus de huit ans après les faits, l’immeuble où un marchand de sommeil hébergeait les terroristes du Bataclan, et qui avait été pris d’assaut par les forces de l’ordre, ne soit toujours pas réhabilité. Nous avons, enfin, consulté les maires la plateforme du Sénat pour mieux comprendre leurs attentes. L’ensemble de ces travaux ont conduit la commission à améliorer le texte et à y introduire de nouveaux moyens d’action pour les collectivités, quelle que soit leur taille.

en un grand texte contre la crise du logement. On peut même parler de rendez vous manqué. Ce n’est que trois mois après avoir déposé ce texte, en décembre dernier, que le Gouvernement semble commencer à prendre la mesure de la crise du logement. Au manque de moyens des élus face à la spéculation foncière s’ajoute le risque de sortie du marché d’un très grand nombre de logements locatifs, faute d’avoir pris à temps les mesures à la hauteur de l’enjeu pour accompagner les bailleurs dans la rénovation de leur bien. Cette impréparation est d’autant plus frappante que, alors même que Christophe Béchu présentait dans la presse de futurs amendements, pourtant en dehors du périmètre du texte examiné, Bruno Le Maire annonçait 1 milliard de coupes budgétaires dans les aides de MaPrimeRénov’. pour le moins incohérentes, les maires n’ont de cesse de demander une solution pour traiter les biens sans maître ou en état d’abandon : 90 % des maires interrogés l’ont évoqué lors de notre consultation. L’habitat dégradé

touchant principalement quelques grandes opérations n’est pas non plus la grande loi de simplification des codes de l’urbanisme ou de la construction et de l’habitation que de nombreux professionnels attendent

à simplifier non pas des dispositifs spécifiques, mais la règle générale ? Monsieur le ministre, fort de l’expérience acquise avec les jeux Olympiques, Notre Dame de Paris

en vous encourageant à faire de tout le territoire national un territoire d’accélération et de simplification pour relancer la construction et donner un logement à l’ensemble à l’ensemble des Français. Le texte que nous voterons cette semaine sera utile, mais nous avons besoin, vous le savez, d’un grand texte sur le logement. Nos concitoyens, nos élus en ont besoin. Mieux, nous avons besoin d’une vision d’ensemble, de cohérence et de long terme, c’est à dire d’une politique du logement qui ne se

concitoyens n’arrivent pas, par manque de volonté et de moyens, ou simplement à cause de procédures trop complexes, à préserver leurs habitats, qui finissent par se dégrader de manière irréversible ?

nous devons préserver nos terres, lutter contre le changement climatique, endiguer la crise économique et financière. Nous devons adapter nos villes et villages aux mouvements des Français entre nos territoires,

Nous devons travailler à ce que l’offre et la demande de logements se rencontrent. Il faut aménager et réaménager notre territoire en conséquence. Cela prendra du temps et aura un coût certain.

du texte a ainsi triplé depuis sa présentation par le Gouvernement, que je sais volontaire sur ce sujet. Le nombre d’amendements déposés à l’Assemblée nationale et au Sénat est la preuve d’une importante mobilisation des élus.

Ma longue expérience de maire me permet d’appréhender sous un certain angle le sujet de l’habitat dégradé et des opérations d’aménagement. Je comprends aussi les besoins des collectivités territoriales, qui fondent beaucoup d’espoirs dans ce texte. Ces problématiques concernent l’ensemble des territoires. Ces collectivités ne pourront continuer à se développer que si nous les aidons à nettoyer – j’insiste sur ce terme, même s’il n’est

Concernant les procédures d’expropriation des immeubles insalubres, le texte, en offrant une possibilité d’action bien plus en amont, semble aller dans le bon sens, tout comme les clarifications introduites en commission. Il faut essayer de prévenir au maximum afin d’éviter les situations irrémédiables. Il en va de même pour les mécanismes relatifs au relogement de personnes et pour ceux qui portent sur la gestion de situations irrégulières

fragiles. Ainsi, des centaines de milliers de personnes se trouvent condamnées à vivre dans des logements vétustes et insalubres. Agir contre la dégradation des copropriétés dans nos métropoles et nos petites villes doit être notre priorité, à la fois pour augmenter le nombre de logements disponibles entrer dans une dynamique d’adaptation de l’habitat à la transition écologique et énergétique. Michèle Lutz et Mathieu Hanotin ont largement guidé, par leur connaissance pointue du terrain, la construction technique de ce texte. Grâce aux propositions concrètes et au travail de nos rapporteures Amel Gacquerre et Françoise Dumont, les collectivités territoriales devraient désormais disposer d’une boîte à outils renforçant la faculté des communes, des intercommunalités et de leurs opérateurs à mener leurs projets. Ce texte aborde, de manière concrète, un sujet crucial pour le bien être et la dignité des Français. Des mesures financières et administratives, encore à nuancer, sont nécessaires pour surmonter les obstacles et permettre d’entreprendre des travaux majeurs. Plus tôt ces actions seront mises en œuvre pour rendre les habitations décentes et respectueuses des normes environnementales de base, moins cher elles coûteront aux propriétaires, aux locataires et aux collectivités. En somme, tout le monde sera gagnant ! Trois points de ce projet de loi ont particulièrement attiré mon attention.

Je salue les ajouts de la commission, qui ont permis d’encadrer ce dispositif tout en le rendant plus souple. Deuxièmement, pour anticiper, prévenir et résoudre les problèmes rencontrés, les pouvoirs publics et les syndics doivent, plus que jamais,

Ainsi, les pouvoirs du maire se trouvent renforcés par la sécurisation du cadre juridique des expropriations nécessaires à la sécurité des citoyens et indispensables au recyclage des habitats urbains. Il en va de même pour l’application des mesures de démolition des constructions jugées irrégulières et présentant des risques pour la sécurité et la santé des résidents. En outre, pour mieux prendre en compte les problématiques des villes moyennes, nous devons porter une plus grande attention aux aux petites copropriétés des centres villes anciens. Ainsi, en permettant au maire de faire procéder d’office à un diagnostic structurel des immeubles en zone d’habitat dégradé, on offre la possibilité d’agir avant que la situation ne devienne irrémédiable. la question du relogement doit, elle aussi, être au cœur de nos préoccupations. Qu’il s’effectue à titre temporaire ou définitif, le relogement de centaines de ménages n’est jamais une opération aisée et représente un frein à la rénovation des copropriétés dégradées.

Anticiper, accélérer, protéger : tels sont les trois axes qui ressortent de ce texte et en font un premier pas technique important. Pour cette raison, nous le voterons. Cependant, monsieur le ministre, votre prédécesseur nous avait promis une grande loi, qui tarde grandement à venir. En parallèle, le Premier ministre a annoncé que le logement serait une des trois priorités de ses cent premiers jours. La boîte à outils aussi pertinente soit elle, ne répond que très partiellement à l’urgence de la crise du logement. Nous attendons davantage ! La parole

Taher Hedfi, Julien Lalonde, Fabien Lavieille, Pape Niasse, Ouloume Said Hassani, Mohamed Cherif Zemar : ce sont les noms des huit victimes de l’effondrement, le 5 novembre 2018, de deux immeubles de la rue d’Aubagne, à Marseille. vous le savez, l’habitat indigne tue ! Cette catastrophe a profondément marqué notre mémoire collective. Avec mon collègue Guy Benarroche, nous avons auditionné les familles et le collectif du 5 novembre Noailles en colère. Une volonté commune a été clairement exprimée : éviter de nouvelles tragédies. Or que s’est il passé après ce drame ? D’autres drames, monsieur le ministre Il y a quatre semaines, un enfant de 7 ans a trouvé la mort dans un incendie survenu à Marseille, dans un immeuble dit « en bon état », mais un logement jugé, lui, « dégradé

vous, que faites vous ? Pas plus tard que cette semaine, vous annoncez 736,8 millions d’euros de coupes budgétaires sur la mission « Cohésion des territoires », dont 300 millions d’euros pris sur l’aide à l’accès au logement et 359 millions au programme « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Seulement 93 000 logements sociaux ont été financés en 2023 ; mais vous, vous détricotez la loi SRU ! Plus de 3 000 personnes, dont 900 enfants, demandent un hébergement à Paris ; mais vous, vous détricotez la loi SRU ! Enfin, 72 % des ménages franciliens peuvent prétendre à un logement très social ; mais vous, que faites vous ? Vous faites la promotion du logement intermédiaire, qui répond aux problématiques de seulement 3 % des demandeurs actuels. Vous l’aurez compris, sur la question du logement, nous ne sommes pas d’accord ! Pourtant, sur ce projet de loi, nous pouvons l’être ; je peux même dire que, globalement, nous le sommes. La puissance publique se mobilise enfin, avec les élus locaux, qui agissent tant bien que mal, comme ils peuvent, mais toujours de leur mieux, avec les outils et les moyens qu’ils ont le rapport de Michèle Lutz et Mathieu Hanotin en est une belle illustration –, et avec les élus nationaux, qui travaillent avec sérieux sur ces sujets prioritaires. C’est un point de convergence entre nous, quelle que soit notre Oui, nous partageons tous le constat alarmant qu’a fait la Fondation Abbé Pierre dans son dernier rapport : « L’écart [est] abyssal entre le nombre de logements indignes et le nombre de procédures engagées. Aussi, l’accélération proposée dans ce projet de loi est plus que bienvenue. Oui, il fallait accélérer ; vous le faites, nous le faisons avec vous. Nous avons amendé et enrichi ce texte, pour qu’il intègre les bailleurs sociaux et pas uniquement les propriétaires privés, pour qu’il soit plus ambitieux en matière de protection des locataires et des propriétaires occupants, ou encore de lutte contre les marchands de sommeil, pour qu’il soit encore plus adapté au fonctionnement des syndicats de copropriétaires,

dans un esprit de recherche de convergence. C’est pourquoi, monsieur le ministre, je compte sur vous pour étudier, voire accepter, sans posture idéologique, les amendements que les écologistes défendront. Par une telle convergence, nous retrouverons l’honneur de la politique, en respectant les millions de ménages, propriétaires occupants ou locataires,

aujourd’hui, face à une crise du logement qui ébranle les fondations de notre société, c’est un message d’urgence que notre groupe tient à porter. qui condamne 330 000 personnes à l’errance sans domicile et plonge 15 millions de personnes dans une précarité alarmante dans un pays aussi avancé que le nôtre, est intolérable. Il y a tant à faire : dans le logement social, pour répondre aux 2,6 millions de demandeurs en attente ; dans la rénovation énergétique, pour rénover les 5 millions de logements mal isolés ; dans la construction, pour relancer un secteur à l’arrêt. Pendant trop longtemps, les mesures prises pour répondre à cette crise ont été insuffisantes, voire contre productives. Nous avons assisté à une libéralisation du secteur du logement

Le 1 février dernier, j’étais à la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Soixante dix ans après cet appel historique, qui avait déclenché un sursaut des citoyens et des pouvoirs publics, nous avons eu droit à un passage éclair du ministre de la transition écologique, qui en a profité pour accabler les sans papiers, qui seraient responsables de leur maintien à la rue et engorgeraient les places d’hébergement. Aucune annonce, aucun sursaut ! Tous ces signaux doivent être perçus pour ce qu’ils sont des attaques contre le droit au logement. Or ces attaques fonctionnent, puisque le nombre de mal logés n’a jamais été aussi élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Victor Hugo l’avait ainsi exprimé en son temps Vous n’avez rien fait tant que le peuple souffre ! Vous n’avez rien fait tant qu’il y a au dessous de vous une partie du peuple qui désespère ! » Aujourd’hui, la souffrance du peuple est là. Elle nous oblige, car c’est un enjeu de dignité humaine. Après avoir allumé le feu, le Gouvernement veut enfiler son costume de pompier et tenter d’éteindre, avec un petit extincteur, un brasier qui devrait mobiliser tous nos canadairs. Le projet de loi qui nous est présenté est intéressant, mais certainement insuffisant. Il a déjà été, il faut le dire, amélioré par l’Assemblée nationale, ainsi que par notre commission des affaires économiques. Je compte sur la séance publique et nos amendements pour lui apporter des améliorations supplémentaires.

et d’intervention sur le bâti, avec une attention particulière portée aux résidents, et des peines plus lourdes contre les marchands de sommeil. Une plus grande vigilance et une fermeté accrue à l’égard des syndics défaillants sont aussi indispensables ; plusieurs de nos amendements visent à aller dans ce sens. Ce texte exprime des intentions louables, qui laissent penser que dans quelques années l’habitat dégradé sera derrière nous. Pourtant, la marche est haute, et l’ascenseur semble toujours en panne : 9 milliards d’euros de travaux seraient nécessaires, selon la Banque des territoires, mais le projet de loi est muet sur les moyens budgétaires mis à disposition pour intervenir. Il y aura bien des prêts collectifs pour les copropriétaires, mais avec quel argent ? Il y aura peut être des interventions publiques, mais avec quels moyens ? Il y aura sans doute davantage de procédures contre les marchands de sommeil, mais avec quels effectifs dans les tribunaux judiciaires ? Il y a quelques jours, vous avez annoncé 10 milliards d’euros d’économies sur le budget de l’État, dont 1 milliard pris sur MaPrimeRénov’. Le nouveau ministre du logement a, quant à lui, prévu de contourner la loi Climat et résilience en modifiant les critères du diagnostic de performance énergétique, laissant ainsi perdurer les passoires thermiques. Alors, avec tout cela, qui ira dire aux mal logés qu’ils peuvent attendre pour avoir un toit sur leur tête, pour allumer le chauffage sans se ruiner, ou pour vivre sans la crainte de voir leur balcon tomber sous leurs pieds Trop de catastrophes sont déjà connues, à Marseille, à Paris, à Lille, ou encore à Grigny, avec la mort de la petite Solange dans l’incendie d’un logement indigne. La difficulté du quotidien, pour les 1,2 million de personnes qui vivent dans une copropriété dégradée, réduites à se dire que, au milieu des moisissures, sous des plafonds qui s’effritent avant, peut être, de s’effondrer, on est déjà mieux qu’à la rue. Nous espérons pouvoir voter ce projet de loi à l’issue des débats qui s’ouvrent. Nous prendrons nos responsabilités et nous souhaitons que le Gouvernement prenne les siennes, en donnant, enfin, des moyens pour répondre à cette crise du logement.

La qualité de cet habitat doit être une priorité de notre action politique. Pourtant, l’habitat dégradé est un phénomène silencieux et massif, encore largement méconnu, qui n’est pas le problème de quelques villes pauvres ou quartiers prioritaires. Je souhaite à cet égard saluer l’initiative de notre assemblée, qui a mis en œuvre une consultation des élus locaux sur la lutte contre l’habitat dégradé afin de mieux connaître les besoins de nos maires et leurs difficultés, et de recueillir leur avis et leurs suggestions sur les principales dispositions de ce texte.

58 % des maires interrogés ont ainsi déclaré avoir une ou plusieurs copropriétés dégradées dans leur commune. Deux tiers d’entre eux estiment que c’est une question importante, voire très importante. Les copropriétés se retrouvent souvent en difficulté et se dégradent au point de nécessiter l’intervention des pouvoirs publics. Leur rénovation est freinée par des difficultés inhérentes à l’habitat collectif, comme le coût élevé des travaux, l’impossibilité d’obtenir le soutien d’une majorité des copropriétaires ou la concentration d’une population défavorisée dans certaines copropriétés. Dans les grands ensembles, dans certains quartiers prioritaires ou dans des centres villes anciens, ce problème peut prendre des proportions très importantes. De lourds moyens financiers et juridiques sont alors

Les copropriétaires paupérisés se retrouvent alors dans l’impossibilité de payer leurs charges ou les travaux d’entretien, tandis que la valeur marchande des immeubles qui se dégradent ne cesse de baisser. Quant aux occupants, ils sont dans l’impossibilité financière de se loger ailleurs. Tous les ingrédients sont donc réunis pour créer de l’habitat indigne, dont un million de Français sont aujourd’hui victimes. Pour nos concitoyens le mal logement peut avoir de réels effets sur la santé, l’éducation, l’équilibre familial, l’insertion sociale et la vie professionnelle. Nous attendons donc beaucoup de ce projet de loi : il faut redonner de la dignité aux personnes, il faut qu’elles puissent vivre dans des logements décents. Je ferai plusieurs observations sur le projet de loi en lui même. S’agissant, tout d’abord, de l’intervention des collectivités et des opérateurs afin de lutter contre l’habitat indigne, je salue les travaux réalisés en commission pour leur donner, légitimement, des outils plus efficaces et plus rapides en vue de permettre une intervention plus précoce des pouvoirs publics, de la rendre moins coûteuse, mieux planifiée, et avec des relogements mieux anticipés et davantage inscrits dans le projet urbain. Je pense ici au syndic d’intérêt collectif et à l’emprunt global et collectif. Néanmoins, j’attends désormais que le Gouvernement s’engage à financer ce dernier, si nous ne voulons pas qu’il reste lettre morte. Par ailleurs, nous relevons sur le terrain que les occupants de logement insalubre sont trop souvent laissés dans l’ignorance des procédures de rénovation et des actes qui les concernent. Pour encore plus d’efficacité et d’opérabilité, le groupe du RDSE a déposé des amendements visant à mieux accompagner, protéger et informer les occupants de ces logements. J’entends ici exprimer notre volonté de simplifier l’accès à l’information des copropriétaires, en posant la dématérialisation comme principe, ou à communiquer le constat d’insalubrité aux copropriétaires en même temps S’agissant de la problématique des marchands de sommeil, nous saluons le travail effectué en commission. Celle ci s’est fondée sur le retour d’expérience des maires pour retenir, à titre préventif, plusieurs évolutions sur le permis de louer et le permis de diviser, facilitant ainsi leurs conditions de mise en œuvre et la lutte contre ces marchands de sommeil. un point de vigilance concernant la procédure d’expropriation. Le nouvel outil envisagé est intéressant ; néanmoins, il ne résout pas l’un des plus gros points de blocage possible lors de la mise en place d’une telle procédure, à savoir celui du relogement des occupants, que ce soit à titre temporaire ou définitif, notamment dans les très grandes opérations, qui nécessitent le relogement simultané de centaines de ménages, principalement dans un parc social déjà saturé. Il s’agit d’un vrai frein pour certaines opérations ; d’ailleurs, plus de 90 % des maires ayant répondu à la consultation ont soulevé cette difficulté, y compris pour des opérations plus ponctuelles.

En la matière, force est de constater que nous devons accélérer et simplifier. Tel est bien l’esprit de ce projet de loi. Face au nombre croissant de copropriétés particulièrement fragiles et à la complexité des procédures, il nous appartient de faciliter de simplifier la vie des acteurs de terrain, à commencer par nos élus locaux. Grâce à ce projet de loi, les élus disposeront demain de nouvelles attributions bienvenues, leur permettant d’intervenir le plus en amont possible sur le bâti dégradé, afin d’éviter de multiplier les constructions délaissées. L’objectif est clair plus de prévention, pour moins de dégradations. Alors, comment les élus pourront ils concrètement agir ? D’abord, en cas d’urgence, lorsque des travaux entrepris engendrent des installations présentant un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, et lorsque la mise en demeure sera restée sans effet, le maire pourra désormais procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites aux frais du propriétaire. Cela va dans le bon sens : il n’est pas juste de laisser une personne en irrégularité exemptée de toute obligation. Les maires pourront également s’appuyer sur un rapport des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) pour motiver leurs arrêtés de mise en sécurité. Je pense également au fait de rendre destinataires du procès verbal de l’assemblée générale de copropriété le maire,

je pense à des professionnels de l’immobilier, mais aussi à des propriétaires. Il est donc logique que les maires et les préfets puissent être présents et participer à ces moments décisifs dans la vie d’une copropriété dont le bâti s’est dégradé. Cela permettra aux acteurs de terrain d’être informés des situations territoriales afin d’agir le plus rapidement possible. Ensuite, mes chers collègues, pour faire davantage de prévention, encore faut il avoir réalisé le bon diagnostic du bâtiment. En ce sens, l’article 8 apporte une solution. ou intercommunal (PLU ou PLUi), des secteurs dans lesquels la réalisation d’un diagnostic global de structure sera obligatoire, une fois tous les dix ans, afin de mieux surveiller la dégradation du bâti et de pouvoir intervenir sans attendre une dégradation irrémédiable. Je crois que nous pouvons saluer ces mesures, qui démontrent que le Gouvernement souhaite faire davantage confiance aux élus locaux en matière de simplification. Mais les élus locaux ne sont pas les seuls acteurs de terrain. N’oublions pas, en effet, le rôle essentiel des copropriétaires, qui demandent, eux aussi, plus d’accompagnement, notamment pour la rénovation énergétique. Or, si nous voulons réduire le nombre de copropriétés dégradées, nous devons faciliter la rénovation énergétique de tous les bâtiments. Cependant, ces travaux souvent très onéreux nécessitent, la plupart du temps, l’octroi d’un prêt. Grâce à l’article 2 du projet de loi, un nouveau type de prêt collectif sera créé pour les copropriétés, qui pourront désormais souscrire un tel prêt pour financer les travaux essentiels à la rénovation énergétique. Afin d’éviter les blocages, il est prévu que tout copropriétaire n’indiquant pas son refus de souscrire un emprunt sera supposé y adhérer.

aux éco prêts à taux zéro (éco PTZ) souscrits au nom des syndicats de copropriétaires. Mes chers collègues, ce texte permettra également de renforcer notre lutte contre un fléau qui gâche le quotidien de nombreux Français, celui des marchands de sommeil. toujours en matière de prévention, il me semble que ce texte met une solution pertinente à la main des collectivités pour anticiper les situations critiques et ainsi mieux protéger les habitants. Je fais référence à la création d’une nouvelle procédure d’expropriation des immeubles qui sont dans un état de dégradation encore remédiable. Aujourd’hui, l’expropriation de certains immeubles insalubres est certes possible, mais elle ne peut être mise en place que pour les immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement d’insalubrité ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’y habiter. Pour que l’expropriation s’applique, il faudra désormais que deux arrêtés de sécurité ou de salubrité aient été pris en l’espace de dix ans sans que les travaux prescrits aient été exécutés. N’oublions pas non plus la réalisation d’un plan de relogement lorsqu’une interdiction temporaire d’habiter d’habiter est prononcée. Avec cette nouvelle procédure, nous ferons davantage de prévention pour éviter les dégradations irréversibles imposant des démolitions coûteuses. Nous éviterons surtout aux habitants le traumatisme d’un départ forcé de leur domicile, tout en économisant l’argent public et en renforçant l’efficacité de l’action de la puissance publique. la lutte contre les marchands de sommeil nécessite également de renforcer les sanctions. Je salue en ce sens les mesures adoptées en commission visant à porter de dix à quinze ans la durée de l’interdiction d’acquisition d’un bien immobilier encourue par un marchand de sommeil.

de déclaration de mise en location ou à faciliter la sortie des indivisions en outre mer. Mes chers collègues, nos concitoyens attendent des mesures fortes en matière de logement. Avant que de futurs textes ne soient soumis au Parlement, nous avons aujourd’hui l’occasion de légiférer sur un enjeu essentiel pour nombre de Français, à savoir la rénovation du bâti dégradé.

il serait difficile de contester la nécessité de faire du chantier des copropriétés dégradées une cause nationale. Les chiffres parlent d’eux mêmes : on compte près de 400 000 logements indignes en métropole – la moitié sont occupés par leur propriétaire – et près de 150 000

Ainsi, dans la loi de 2014, plusieurs mesures ont déjà renforcé l’arsenal législatif en la matière, mais force est de constater qu’elles demeurent insuffisantes. En tant que législateur, il était donc de notre devoir de doter au plus vite les collectivités de moyens supplémentaires et renforcés pour lutter contre ce phénomène, qui menace notre cohésion sociale. Je tiens à saluer le travail de Mme la rapporteure, qui a simplifié et amélioré ce texte dans un temps très contraint. Les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain l’ont aussi amélioré en commission. Mme la rapporteure d’avoir tenu compte de nos amendements, particulièrement de ceux qui ont pour objet les aides aux collectivités. En effet, en prenant appui sur le rapport de Mathieu Hanotin, maire de Saint Denis, et de Michèle Lutz, maire de Mulhouse, nous avions en tête trois objectifs

introduisant le transfert de la compétence pour le recouvrement des amendes relatives au permis de louer aux communes et aux EPCI. Par ailleurs, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Nous avons également instauré un droit au relogement pérenne pour les occupants qui ne pourront pas réintégrer leur habitat initial, et une obligation de relogement définitif, si les travaux ne sont pas réalisés. Nous avons introduit une sanction en cas de refus d’établir un bail écrit ou de remettre une quittance. Nous avons également élargi les mesures de protection des occupants dès le début de la procédure contradictoire contre des menaces ou congés abusifs de la part de propriétaires. l’ajout de la rénovation de l’habitat dégradé dans les missions de l’ANCT pour mieux accompagner les maires qui ne disposent pas de l’ingénierie nécessaire pour intervenir dans les petites copropriétés. Je pense également à l’extension à quinze ans de l’interdiction d’acquisition d’un bien immobilier qui est encourue par un marchand de sommeil.

Les débats qui s’ouvrent aujourd’hui nous permettront donc, je l’espère, de perfectionner encore ce texte, qui va dans le bon sens. La parole

Oui, libérer le logement est possible. Cela passe par une nouvelle donne, un volontarisme politique, qui octroie aux maires les moyens de mener une véritable politique d’aménagement du territoire. Le texte qui nous est présenté cet après midi est technique. Il n’est qu’un volet infime des moyens nécessaires que l’on doit donner aux élus locaux pour essayer de ralentir effectivement la dégradation de l’état de santé du logement en France. Il faut donc aller plus loin,

les schémas départementaux du logement. Il faut les généraliser ! L’État octroie des moyens, sous l’autorité des préfets – ils sont indispensables –, avec les conseils départementaux et avec les élus locaux, pour écrire une nouvelle page de l’histoire du logement dans notre pays. Toutes les initiatives

Deux mesures sont à prendre. D’abord, créer un véritable choc de l’offre, alors que plus de 150 000 logements par an manquent pour répondre à la demande. Ensuite, permettre à chacun de rénover des logements existants grâce à un calendrier raisonnable. C’est pour relever ce deuxième défi que vous présentez le projet de loi que nous examinons aujourd’hui, monsieur le ministre. Une part prépondérante du parc de logements dégradés correspond aux immeubles d’habitation collective. Parmi ces passoires thermiques, nombreuses sont celles qui relèvent de la copropriété privée. du groupe Union Centriste saluent le plan Initiative Copropriétés, piloté par l’Anah, qui propose un accompagnement, afin de requalifier plus de 80 000 logements situés dans des copropriétés. Voilà une initiative salvatrice Mais ce n’est pas suffisant, mes chers collègues. Alors que les occupants sont parfois dans des locaux insalubres, voire dangereux, la complexité du droit ressemble beaucoup au mystère de la pierre de Rosette. Chacun a pu noter la technicité du texte qui nous est présenté, et ses propositions de bon sens également. On sent pleinement la patte de Michèle Lutz et de Mathieu Hanotin, deux élus locaux ayant une profonde connaissance du terrain. Nos rapporteures, Mmes Amel Gacquerre et Françoise Dumont, se sont pleinement investies pour enrichir le texte, afin d’en faire un véritable outil d’accélération de la rénovation des habitats indignes et dégradés. Je souhaite saluer trois mesures introduites, qui me semblent être fondamentales pour donner aux élus et à l’État les outils pour atteindre cet objectif. Tout d’abord, la possibilité pour toutes les copropriétés de souscrire un prêt collectif pour le financement de travaux essentiels et de rénovation énergétique. C’est un pas en avant pour que les propriétaires les plus modestes puissent s’associer pour financer des travaux. En commission, sur l’initiative de notre rapporteure Amel Gacquerre, les modalités de mise en œuvre de ce prêt ont été assouplies.

Cette mesure permettra de sécuriser le traitement de celles dont la gestion a été confiée par le juge à un tiers. Elle permettra également d’éviter la saisie des fonds publics par les créanciers tout en assurant leur bon emploi. Enfin, nous avons renforcé la place des communes dans le processus de rénovation. Le nouvel article 2 A permettra ainsi aux communes d’être compétentes en matière de permis de louer, même lorsqu’elles n’ont pas la compétence L’article 7 A transfère également la compétence pour le recouvrement des amendes relatives au permis de louer aux communes et aux EPCI compétents. Nos collectivités doivent bénéficier d’un arsenal complet en matière de location pour assister les copropriétaires souhaitant rénover leur habitation.

non plus de logements proposés à des prix ou loyers qui soient abordables et adaptés au pouvoir d’achat de nos concitoyens ! Et il y a trop de passoires thermiques, alors qu’il nous faut réduire drastiquement les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre

C’est là un enjeu de taille et un combat de longue haleine. Année après année, avec la loi Alur de 2014 ou d’autres textes, l’arsenal législatif et réglementaire français s’est renforcé en la matière. Pourtant, régulièrement encore, dans nos villes, des hommes, des femmes, des enfants souffrent, voire perdent la vie du fait d’un habitat dégradé non rénové.

C’est pourquoi nous voterons l’essentiel des dispositions de ce projet de loi. Mais nous proposons aussi d’aller plus loin dans la lutte contre l’habitat dégradé. Ainsi, largement inspirés de nos discussions avec des collectivités et des associations, nos amendements vont dans l’intérêt des élus locaux, mais aussi des occupants à protéger. Par exemple, nous souhaitons, à l’article 3, renforcer l’effectivité de l’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable, en la faisant mieux coller à la réalité des arrêtés pris par les maires.

C’est pourquoi nous souhaitons, comme le prévoyait l’article 3 A, non seulement que l’expérimentation d’expropriation des parties communes prévue par la loi Alur soit prolongée, mais surtout qu’elle devienne possible pour les organismes de foncier solidaire Plusieurs d’entre eux ont travaillé des projets concrets en ce sens ; ce serait leur envoyer un très mauvais signal que de les empêcher de faire ce test. Dans le même esprit, nous soutiendrons la possibilité pour les organismes d’HLM d’utiliser un bail réel solidaire d’activité. Enfin, vous vous en souvenez sûrement, ma ville de Lille a été touchée en novembre 2022 par un drame lié à l’habitat : deux immeubles se sont effondrés soudainement rue Pierre Mauroy, coûtant malheureusement la vie à l’un des occupants. Sans la présence d’esprit de jeunes riverains, peut être que le bilan aurait même été plus lourd. La particularité de ce drame est qu’il n’est pas un drame de l’habitat indigne ou insalubre et que les occupants n’étaient ni victimes de marchands de sommeil ni particulièrement paupérisés. C’est pourquoi nous soutenons l’article 8, qui introduit l’obligation d’un diagnostic structurel régulier pour les immeubles de certains secteurs d’habitat dégradé. Et nous souhaitons le compléter par un amendement tendant à autoriser les collectivités à cibler les secteurs d’habitat dégradé, mais aussi les centres anciens qui abritent des immeubles des siècles passés.

En témoignent les textes de loi adoptés ces dernières années dans ce domaine : la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la loi Alur de 2014, la loi Élan de 2018. Toutes ont doté les pouvoirs publics de moyens supplémentaires pour réduire la mise en location de logements indignes et l’activité de marchands de sommeil. On pourrait ajouter le plan Initiative Copropriétés, lancé en 2018 par le Gouvernement ou encore l’ordonnance de septembre 2020, qui a permis la refonte des polices administratives spéciales de lutte contre l’habitat indigne et un partage plus clair des compétences entre le préfet et les maires. Pour autant, la situation demeure toujours aussi préoccupante. Le rapport Hanotin Lutz a évalué à 400 000 le nombre de logements indignes et à 100 000 le nombre de copropriétés fragiles. Cette situation a été confirmée par la consultation réalisée par notre présidente et notre rapporteure auprès des maires. Leur attente est très claire : garder la main sur le sujet de l’habitat dégradé, en collaboration avec l’État. Toutefois, ils déplorent un manque d’information, notamment en provenance du registre national d’immatriculation des copropriétés ou encore de l’Anah, une complexification des procédures ou la méconnaissance de certains outils comme le plan Initiative Copropriétés ou les opérations d’intérêt national. Au milieu de ces lacunes, seules les opérations de restauration immobilière semblent faire consensus en matière de procédures. Avec une constante, ils regrettent tous, ou en tout cas très largement, la difficulté de reloger les habitants concernés. Dans ce contexte, l’objet du projet de loi, à savoir simplifier les procédures judiciaires et administratives pour accélérer le travail de copropriétés les plus dégradées, Il s’agit en fait d’intervenir le plus tôt possible avant que l’habitat dégradé ne devienne indigne, c’est à dire qu’il ne soit susceptible d’être démoli. Il s’agit aussi de préserver l’intégrité des bâtiments et de réduire le coût sur le long terme. En ce sens, plusieurs dispositifs contenus dans le texte sont tout tout à fait opportuns. En matière de prévention, il est envisagé de créer une nouvelle procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des propriétaires de logements frappés de péril ou d’insalubrité. Le droit de préemption simplifié devrait permettre, à la demande des collectivités, de réaliser des actions nécessaires à un office public de l’habitat (OPH), un plan de sauvegarde ou une opération de requalification de copropriétés dégradées. L’expropriation pourrait ainsi devenir possible avant que la situation ne soit devenue irrémédiable. ne soit devenue irrémédiable. Le projet de loi prévoit aussi la possibilité pour les copropriétés de souscrire un prêt bancaire collectif pour faciliter le financement de travaux d’entretien et de préservation essentiels. Une garantie publique pour les copropriétés, dont la situation financière est dégradée, a également été ajoutée. En revanche, que se passera t il dans le cas où pour les autres copropriétés, l’un ou plusieurs de ses membres deviendraient défaillants lors de la période de remboursement ? Qui prendra la relève ? Et surtout, avec quels financements ? Afin d’aider les petites communes à mieux prévenir les phénomènes d’habitat dégradé, la commission a

La commission a tenu aussi à apporter plus de souplesse à un dispositif trop rigide, notamment en créant un label attestant de compétences utiles au traitement des difficultés financières. Le texte prévoit enfin la possibilité pour les opérations de demander la scission de grands ensembles en copropriété pour faciliter la gestion et éviter les dégradations de biens. D’autres éléments, notamment en matière pénale, visent à sanctionner les marchands de sommeil, je n’y reviendrai pas.

permettant ainsi un développement foncier cohérent avec les modalités d’intervention de l’association. Quel est l’avis de la commission ? Comme cet amendement

Bernard Buis. Cet amendement de mon collègue Didier Rambaud vise à supprimer une disposition introduite à l’article 26 4 de la loi du 10 juillet 1965 par la loi de finances pour 2024 permettant la souscription d’un éco PTZ au nom au nom du syndicat de copropriétaires à la même majorité que celle qui est requise pour le vote des travaux, au profit de la nouvelle formule d’emprunt qui reproduit ces conditions.

faciliter le préfinancement des subventions publiques. Ces prêts ont vocation à bénéficier d’une garantie publique dans les copropriétés en difficulté. Il nous paraît donc important de préciser dans la loi que le remboursement anticipé du solde de l’emprunt à la suite du versement des subventions publiques ne donne lieu à aucuns frais ni indemnité. Nous profitons de cet amendement pour demander au Gouvernement de reconsidérer la recommandation de la Banque des territoires considéré à 150 millions d’euros par an pour permettre au réseau Procivis d’avancer sans intérêt le montant des subventions publiques.

L’idée de fixer la durée du prêt par décret et de retenir une durée unique résulte du rapport de la Banque des territoires : celle ci avait estimé que la durée du prêt devrait être suffisamment longue pour minimiser les charges

L’amendement n° 84 vise à aller au delà des facilités de remboursement anticipé prévues par le texte en proposant un remboursement sans frais.

pour que soit requis l’accord de la banque et du garant avant le transfert au nouveau propriétaire de la charge de la contribution au remboursement de l’emprunt. L’amendement tend à rétablir le principe d’un transfert

Sénat l’a réintroduite dans la forme existante pour les autres prêts, c’est à dire un remboursement de droit à la vente du lot, sauf accord du prêteur, de la caution et de l’acquéreur. Par son amendement, le Gouvernement propose une formulation

Le nouveau prêt global et collectif créé à l’article 2 ne pourra fonctionner que si les banques et les cautions peuvent acquérir une juste vision du risque et respecter leur obligation de pratiquer un prêt responsable, c’est à dire de ne prêter qu’à

Toutefois, cette consultation ne peut se faire que dans le cadre d’une analyse de solvabilité classique, à l’image de ce qui existe déjà pour les crédits à la consommation et immobiliers. Le dispositif proposé prévoit cette même possibilité pour l’organisme de caution, ce qui entraîne une adaptation des articles 751 2 et suivants du code de la consommation afin de permettre la levée du secret professionnel des agents de la Banque de France à l’égard de ces organismes.

des copropriétaires. La commission a voté un amendement visant à limiter le montant total des fonds empruntés au total des quotes parts des dépenses des copropriétaires qui n’ont pas refusé le prêt.

Dans le cadre du nouvel emprunt créé à l’article 2, tous les copropriétaires participent à l’emprunt selon les modalités contractuelles, ou, en cas de refus, versent dans un délai de six mois la totalité de leur quote part du prix des travaux. L’option d’échelonnement des paiements prévue à l’article 33 doit donc être écartée.

par décret et la différence de durée entre les deux dispositions pourrait rendre la situation très difficile à gérer pour les syndics, voire impossible, si un nombre important de copropriétaires demandaient à en bénéficier. Cette exemption nous semble nécessaire. Aussi la commission émet elle

soutenu et réglementé par l’État, s’inscrivant dans la lignée des PTZ déjà existants et qui favorisent aujourd’hui les emprunteurs des zones urbaines et pour des logements neufs.

L’amendement n° 19 vise à créer un nouveau crédit d’impôt pour le financement à taux zéro des travaux permettant de garantir la salubrité, l’intégrité de l’immeuble ou la sécurité des personnes vivant en copropriété. Un tel dispositif crée un nouveau coût pour l’État. Or il n’a pas été évalué.

pour faire face à un afflux de touristes : le va et vient des valises, la diffusion des codes d’accès et la surutilisation des ascenseurs dégradent bien souvent les parties communes. De plus, il est rare

nous semble particulièrement important en ce qu’il étend le champ d’intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique à l’ensemble des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté.

Plus de 80 000 copropriétés sont considérées comme fragiles, c’est à dire présentent des impayés supérieurs au seuil d’alerte ; elles abritent plus de 4,8 millions de ménages vivant sous le seuil de pauvreté. Or le montant annuel des travaux de rénovation à réaliser, et donc potentiellement à financer, au cours des prochaines années est de l’ordre de 9 milliards d’euros. La garantie publique est, de ce fait, indispensable. Les travaux de la commission ont à juste titre révélé que cette garantie publique n’était pas financée.

de tenir compte de l’élargissement de son champ d’intervention à l’ensemble des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté, au lieu des seuls travaux de rénovation énergétique. Ce fonds étant également mentionné dans le code de l’énergie et dans le code de la consommation, il est nécessaire d’adopter des mesures de coordination tendant à modifier l’intitulé de ce fonds

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Je vous remercie dire combien j’ai été émue d’entendre plusieurs de nos collègues rendre hommage à Claude Dilain, figure importante et emblématique pour les socialistes et pour toute la gauche en Seine Saint Denis. Placer ce projet de loi sous son patronage est un symbole fort. L’article 3 crée un droit d’expropriation pour les immeubles indignes à titre remédiable. Cette mesure correspond à la recommandation n° 1 du rapport Hanotin Lutz, qui préconise de doter la puissance publique d’une capacité à agir en expropriation même lorsque le caractère irrémédiable de la

Cependant, la double condition à laquelle est subordonné, dans le projet de loi, l’engagement de la procédure, à savoir l’absence d’exécution des mesures prescrites par au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité

L’expropriation doit se justifier par un motif d’intérêt général et être précisément encadrée. Pour cette raison, le Conseil d’État a logiquement et fortement insisté, dans l’avis qu’il a rendu sur ce projet de loi, sur la nécessité de prouver une carence persistante du propriétaire ou de la copropriété.

au terme de longs échanges, notamment avec le Conseil d’État, comme l’a rappelé Mme la rapporteure, qui permet de préserver la sécurité juridique du dispositif, lequel porte dès lors une atteinte proportionnée

pour pouvoir enclencher la procédure de l’article 3. En effet, une telle mesure pourrait limiter le caractère opérationnel du dispositif en prescrivant des contraintes inappropriées. Il est du ressort de la nouvelle procédure d’assurer la protection des occupants des logements indignes et l’interdiction d’utiliser des locaux devenus dangereux. Pour autant, cette protection ne va pas au delà d’une telle interdiction d’utiliser. d’utiliser. Les commerçants évincés des locaux dangereux pourront par ailleurs se voir proposer un local de remplacement dans le cadre de la procédure d’indemnisation ultérieure. Quel est l’avis de la commission ? Pour rappel,

être expropriés dans les mêmes conditions que les logements, en particulier pour ce qui est des modalités de fixation des indemnités d’expropriation, qui sont plus avantageuses pour l’expropriant. ce faisant, de faciliter la mise en œuvre de la nouvelle procédure. Il nous semblait également légitime que les occupants de locaux professionnels et commerciaux puissent bénéficier, eux aussi, d’un relogement par l’expropriant. Ces deux amendements visent à supprimer cette obligation de relogement amendements visent à supprimer cette obligation de relogement lorsque les locaux commerciaux et professionnels sont frappés d’une interdiction temporaire d’utiliser, car cette obligation pourrait retarder la mise en œuvre de la procédure d’expropriation

met fin à tous les baux existants sur une parcelle ; autrement dit, les baux s’arrêtent au moment de l’expropriation et les locataires sont protégés et indemnisés. La nouvelle procédure d’expropriation mise en place par ce projet de loi prévoit un transfert des baux existants au moment de l’expropriation aux nouveaux propriétaires, en général une collectivité territoriale ou un opérateur public. Très concrètement, cela signifie que, si l’immeuble exproprié comprend un commerce en rez de chaussée, le bail commercial sera maintenu. Par exemple, si le bail court neuf ans, le commerce pourrait se maintenir neuf ans. Comme l’a très justement souligné ma collègue, les acteurs de la lutte contre l’habitat indigne nous indiquent qu’un tel dispositif pourrait allonger considérablement les délais des opérations de requalification du bâti dégradé et mettre en péril leur équilibre.

autant que possible aux occupants de rester dans leur logement, ce qui n’empêchera pas leur éviction temporaire, si nécessaire, le temps des travaux. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements

puissent être immédiatement saisies. Il est en conséquence prévu de supprimer la mesure de séquestre pour la remplacer par une information systématique du procureur de la République par l’expropriant qui s’apprête à verser des indemnités à une personne mise en cause pour des faits d’habitat indigne. Cette disposition permettra au procureur de la République de procéder à la saisie immédiate de ces sommes

Quel est l’avis de la commission ? Il est vrai que les collectivités hésitent parfois à faire exécuter les travaux d’office sur un bâtiment frappé d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, par crainte de ne pouvoir récupérer les fonds avancés. Cela dit, il est déjà prévu que les frais avancés par la collectivité pour effectuer ces travaux d’office soient récupérés. En effet, le comptable public assure le recouvrement des créances émises, et il lui appartient de poursuivre ce recouvrement par tous moyens à sa disposition, selon les règles applicables du livre des procédures fiscales, y compris la saisie administrative sur les comptes bancaires du propriétaire débiteur ou sur les revenus ou créances de ce dernier sur des tiers. Ces modalités de recouvrement ne sont peut être pas parfaites, mais prévoir une cession gracieuse automatique de l’ensemble du bien, dont le montant excède parfois largement

et où le propriétaire ne s’est pas, au moins en partie, acquitté de sa créance envers elle dans un délai de deux ans, le logement concerné soit automatiquement cédé, à titre gracieux, à ladite commune. C’est un peu radical…

Si le danger est imminent et manifeste, il n’y a en réalité pas besoin de faire procéder à une visite des locaux. Pour rappel, l’article L. 511 19 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’activation de la procédure d’urgence

de danger immédiat, de situation grave et imminente, le maire doit déjà, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et ce au titre de l’article L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales. Il doit notamment procéder à l’évacuation des occupants, instaurer un périmètre de sécurité, prescrire l’exécution des mesures de sécurité nécessaires et appropriées sur un immeuble. Par ailleurs, l’article 122 7 du code pénal protège l’autorité compétente amenée à procéder à une visite en cas de danger imminent et manifeste.

Mme Viviane Artigalas. L’expérience de la gestion de crise des périls et des évacuations montre que les conditions de réintégration ne sont pas toujours satisfaisantes. Des arrêtés d’interdiction d’occuper sont levés dès lors que les périls sont écartés, alors même que le logement ne respecte pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité. Aussi proposons nous, par cet amendement, que les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne prescrivent explicitement les mesures requises afin que le logement, qui était régulièrement occupé, réponde aux normes de confort et d’habitabilité en sortie d’habitat indigne. indigne. Quel est l’avis de la commission ? En commission, nous avons rejeté un amendement similaire, qui visait à permettre d’imposer la mise aux normes de décence

amendement a pour objet de transformer automatiquement l’obligation d’hébergement que doit le propriétaire au locataire, lorsque son logement est frappé d’une interdiction temporaire d’habiter, en obligation de relogement pérenne, dès lors que les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été réalisés dans le délai imparti. Ce délai est trop court, car, lorsque le propriétaire n’achève pas les travaux

est à M. Guy Benarroche. Les drames liés à l’habitat dégradé se multiplient et la question du relogement, nous venons de le voir, est un enjeu clé.

qui ont élaboré une charte destinée à mieux préciser ce qui détermine le caractère adapté du logement ou de l’hébergement qui doit être proposé aux occupants protégés. Il s’agit donc de renforcer la protection des occupants lorsque l’interdiction d’habiter est prononcée à titre définitif et que le propriétaire est tenu d’assurer le relogement.

se situant à proximité du logement d’origine pour permettre aux occupants évincés de poursuivre leur vie personnelle, familiale, professionnelle et scolaire, et adaptée à la composition du foyer et le cas échéant aux personnes en situation de handicap

Mme Viviane Artigalas. Les associations et collectifs réunis dans le mouvement de lutte contre le mal logement à Marseille témoignent que de nombreux occupants en situation de précarité sociale se trouvent également sous le joug de marchands de sommeil. Ils jugent indispensable de lever les obstacles qui entravent la reconnaissance de leur situation et leur protection, afin qu’ils puissent déposer plainte et suivre les procédures de façon sereine. Certains propriétaires indélicats parviennent à obtenir la résiliation judiciaire des baux en raison du défaut de paiement des loyers et des charges. Les occupants sont sont alors privés de leur droit au relogement et, éventuellement, de leur recours en indemnisation. Pour renforcer la protection des occupants, nous proposons d’introduire à l’article 521 1 du code de la construction et de l’habitation une présomption de bonne foi de l’occupant. Ainsi le droit au relogement s’appliquerait il, sauf en cas de mauvaise foi avérée de l’occupant.

Il s’agit d’un principe général du droit des contrats qui se trouve être plutôt protecteur pour les plus vulnérables, puisqu’il vise à prévenir l’abus de droit, y compris les clauses abusives au contrat.

aucune précision n’est donnée quant au délai à l’échéance duquel le terrain devrait être rétrocédé aux propriétaires de l’immeuble ; on ne sait pas non plus précisément ce que recouvre le « droit réel de ré accession » des copropriétaires. Plus fondamentalement, il nous paraît dangereux d’essayer de contourner les difficultés budgétaires d’une copropriété en jouant sur le démembrement de propriété. Cela reviendrait à créer une hypothèque

rectifié. Les agents assermentés du service municipal du logement disposent d’un droit de visite des locaux d’habitation, après accord du propriétaire ou du locataire, ou au besoin après autorisation judiciaire, pour en constater l’état d’occupation. Mais, paradoxalement, ils ne disposent pas d’un droit d’accès de principe aux parties communes des immeubles en copropriété. Cet amendement a pour objet de rendre les contrôles sur place beaucoup plus efficaces, tout en les sécurisant juridiquement actuellement, plusieurs visites sont nécessaires pour accéder à un immeuble, la sollicitation préalable des copropriétaires ou du syndic entraînant des délais considérables et préjudiciables.

Les agents assermentés du service municipal du logement sont habilités à visiter les locaux à usage d’habitation, et non les parties communes. L’accès aux parties communes doit donc leur être ménagé uniquement en tant qu’il leur permet d’accéder

effet, le Gouvernement considère que l’article L. 651 6 du code de la construction et de l’habitation permet aux agents assermentés, qui sont nommés par le maire et prêtent serment devant le juge du tribunal d’instance, de visiter

[s]ans pouvoir opposer le secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle ». Nous proposons d’ajouter que les syndics de copropriété sont également soumis à cette obligation.